Monsieur le président,

Messieurs les ministres, mes chers collègues, madame, c'est- souvenons-nous -avec beaucoup d'émotion de tristesse que nous avons appris, le 27 août dernier, la disparition du doyen de notre assemblée. Philippe Madrelle nous a quittés au terme d'un combat contre la maladie qu'il menait courageusement, en poursuivant ses activités.

de nombreuses personnalités politiques, dont le président de son groupe, le groupe socialiste et républicain, Patrick Kanner. Figure emblématique du département de la Gironde, Philippe Madrelle voua sa vie entière à un engagement inlassable au service de ses compatriotes et de l'intérêt général. Ses grandes facultés d'écoute et d'empathie, son humanisme, son indéfectible esprit de justice, de solidarité et de fraternité étaient unanimement salués et suscitaient le respect de tous. Profondément ancré dans son territoire- oui, « son » territoire ! -, il exerça avec une longévité exceptionnelle, et sans doute inégalée, ses mandats locaux et nationaux. Il fut maire de Carbon-Blanc pendant un quart de siècle, de 1976 à 2001. La confiance des électeurs du canton de Carbon-Blanc, jamais démentie, renouvelée à sept reprises, lui permit de siéger sans discontinuité quarante-sept années durant au sein de l'assemblée départementale. Il présida aux destinées du département de la Gironde pendant jusqu'en 2015, avec une brève interruption de 1985 à 1988. pour la première fois au Sénat en 1980, après douze ans de mandat de député, et ensuite réélu sénateur à quatre reprises, il siégea pendant près de trente-neuf ans dans notre hémicycle. Comme il en convenait lui-même en prenant la parole devant le Sénat, à cette place même, comme doyen d'âge en 2017, « sans doute ne sera-t-il plus possible, à l'avenir, de s'exprimer avec le recul de cinquante années de vie parlementaire ». Et pourtant, ce recul n'est pas inutile, me semble-t-il, à notre vie démocratique ... Philippe Madrelle était né le 21 avril 1937 à Saint-Seurin-de-Cursac, petite commune du Blayais dans le nord de la Gironde, là même où il repose aujourd'hui. Il fut immergé dans la vie politique dès son plus jeune âge. Son père, contrôleur des contributions, était aussi un militant SFIO et un et un élu local, conseiller municipal, puis maire de la commune. Le sport occupa une place importante dans sa jeunesse. Coureur de fond, il fut plusieurs fois champion universitaire de 400 mètres. Ainsi qu'il le déclara plus tard, cette dure école du sport lui donna des leçons de courage, d'endurance, d'humilité et de loyauté. Titulaire d'un baccalauréat de philosophie et d'un certificat d'études littéraires générales de la faculté de Bordeaux, il débuta dans la vie professionnelle comme instituteur dans un village, puis comme professeur d'anglais. Mais Philippe Madrelle fut très tôt attiré par la vie politique, où l'entraînèrent tant ses inclinations personnelles que cette solide tradition de militantisme familial.

Mieux vaut avoir un métier ». De même, son frère Bernard, également enseignant à l'origine, s'orienta ensuite vers la politique et fut longtemps député de la Gironde, de 1978 à 2007. Dès 1965, à l'âge de 28 ans, Philippe Madrelle fut élu conseiller municipal d'Ambarès. Deux ans plus tard, il devint le suppléant du député René Cassagne. Cet ami de son père, autre grande figure du socialisme girondin, fut, selon ses propres dires, « l'inspirateur de toute [sa] carrière ». Philippe Madrelle lui succéda à l'Assemblée nationale en 1968. À l'âge de 31 ans, il fut alors le plus jeune député de France et le benjamin du groupe socialiste. Il ne savait pas encore que le destin le conduirait, cinquante années plus tard, à devenir le doyen du Sénat. Il fut successivement conseiller général en 1969, adjoint au maire de Carbon-Blanc en 1971, puis, comme je l'ai évoqué, maire de cette commune. Quelques mois après son élection comme maire, il devint, à 39 ans, le plus jeune président de conseil général de France. Il s'investit avec passion dans cette fonction. Il s'attacha sans relâche à favoriser le développement de son département- un développement, je souhaite le préciser car c'est un point auquel il tenait par-dessus tout et dont il m'avait entretenu, entretenu, équilibré entre espace urbain et monde rural, entre la métropole bordelaise et les autres composantes du plus vaste département de France Pour ce faire, il dota l'assemblée départementale d'instruments d'action novateurs, comme le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes. Il mit également en place des contrats de développement social, urbain et rural, pour soutenir tant les quartiers sensibles que les zones rurales fragilisées. En 1980, il fit donc son entrée au Sénat. Expliquant son choix de quitter l'Assemblée nationale pour rejoindre notre assemblée, il déclarait alors que sa fonction de président de conseil général l'orientait tout naturellement vers la chambre représentant les collectivités territoriales. En 1981, il succéda à André Labarrère comme président du conseil régional d'Aquitaine. Pendant quelques années, il fut à la fois sénateur, président de conseil général et président de conseil régional

il avait rétorqué qu'il serait prêt à donner l'exemple en cas de vote d'une loi limitant le cumul des mandats, tout en faisant observer que « la carte de visite est imprimée par le [seul] suffrage universel ». Au Au Sénat, Philippe Madrelle choisit de siéger à la commission des affaires étrangères et de la défense, dont il fut membre pendant plus de vingt ans avant de rejoindre la commission de la culture en 2011, puis la commission de l'aménagement du territoire en 2014. C'est donc tout naturellement qu'il prenait régulièrement part aux débats sur les questions de politique étrangère ou de défense. Il avait gardé de sa jeunesse un intérêt particulier pour le milieu sportif et avait à coeur d'intervenir, presque chaque année, sur le budget de la jeunesse et des sports. Il profitait également, le plus souvent possible, des séances de questions orales pour défendre les intérêts de son cher département de la Gironde sur des questions qui lui tenaient à coeur. Philippe Madrelle fut un acteur majeur de la décentralisation en Gironde. Décentralisateur acharné, il était, dans tous les sens du terme, un « Girondin Dès 1980, il déclarait croire profondément en l'avenir de la décentralisation, « cette réforme essentielle pour l'avenir démocratique de notre pays ». Aussi s'engagea-t-il avec conviction en faveur des lois de décentralisation initiées par le président Mitterrand et Gaston Defferre. Il fut en même temps, tout au long de sa carrière politique, un défenseur du monde rural et des collectivités territoriales, du binôme département-communes. Son épouse me disait combien la rencontre avec les maires, jusqu'au dernier instant, était pour lui un moment où il nourrissait son action. il écrivait dans une tribune libre publiée dans : « Comment imaginer de renoncer à l'inestimable atout de proximité que constitue le couple département-communes ? »

En 2014, au cours de la campagne pour les élections sénatoriales, il dénonçait, transgressant même le périmètre établi par sa propre formation politique, la réforme territoriale en cours comme portant atteinte à ce binôme ce binôme département-communes, qui avait permis- je reprends ses mots -de « mettre fin à des siècles de féodalité ». Philippe Madrelle avait pressenti, avant tout autre, le péril mortel que ferait courir à notre démocratie une fracture territoriale qui ne cesse, depuis des années, de s'élargir. Souvenons-nous de son allocution de président d'âge en 2017 : « nous avons tous conscience qu'il y a urgence à prendre en compte la lassitude et les attentes des élus locaux, qui animent dans la proximité les cellules de base de la République et de notre démocratie représentative ». Sa carrière de parlementaire et d'élu local l'avait également convaincu, depuis longtemps, de la nécessité d'une seconde chambre, assurant la représentation de la Nation selon une approche fondée sur les territoires, et ce même s'il pensait que le Sénat devait sans cesse s'adapter et se moderniser.

des régimes démocratiques ». Selon ses propres mots, le Sénat, loin d'être l'assemblée conservatrice parfois décrite par ses détracteurs, était l'assemblée de l'approfondissement du travail législatif, « un lieu de travail serein et sincère, dont la valeur essentielle est le respect : respect des principes de la République, respect du Gouvernement, respect du pluralisme et de la diversité idéologique, et surtout respect des collègues et de leurs expressions ou opinions, en toutes circonstances ». Ces mots, je crois, sont la meilleure présentation du Sénat. Soucieux de la préservation et de la transmission de la mémoire de l'action des sénateurs, Philippe Madrelle a tenu à déposer au Sénat, au début de cette année, son fonds d'archives privées liées à l'exercice de son mandat sénatorial.

un parlementaire estimé, un humaniste. C'est un hommage à un défenseur inlassable de la ruralité et des collectivités territoriales, un acteur majeur de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, un partisan du bicamérisme, et notre doyen- ce qui a un sens pour chacun d'entre nous, quel que soit le groupe dans lequel nous siégeons. À ses anciens collègues des commissions des affaires étrangères, de la culture et de l'aménagement du territoire,

à ses enfants, à toute sa famille et à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je souhaite redire la part que le Sénat prend à leur chagrin. Philippe Madrelle, nous ne l'oublierons pas comme ça, comme le temps qui passe Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame, nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer la mémoire du sénateur Philippe Madrelle. En tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, j'ai témoigné, lors de ses funérailles à Bordeaux, au nom du Gouvernement, de la reconnaissance de la République à l'un de ses plus fidèles serviteurs. Philippe Madrelle aura connu un parcours politique exceptionnel. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le président, lui-même indiquait, lors du discours qu'il prononça comme doyen d'âge du Sénat, à l'ouverture de la séance ayant suivi le dernier renouvellement de la Haute Assemblée, en 2017, que des parcours comme le sien ne seraient bientôt plus possibles. Il aura en effet exercé les mandats de sénateur, député, maire de Carbon-Blanc, président du conseil général de la Gironde et président du conseil régional d'Aquitaine. C'est une vie entière consacrée à la politique et au bien commun Cet engagement tient sans doute à un atavisme paternel. C'est son père Jacques, adhérent de la SFIO et lui-même maire, qui l'éveillera à la politique et au militantisme. Mais il y a une dimension personnelle dans ce parcours hors du commun Philippe Madrelle aimait la politique dans le sens le plus noble du terme, parce qu'il aimait les gens et ne répugnait pas non plus au combat politique- on peut même dire qu'il en avait le goût. Seule la victoire a un intérêt », avait-il confié à son biographe dans la perspective de la publication d'un ouvrage retraçant son parcours. Cette ardeur au combat politique n'était peut-être pas étrangère à son goût pour la compétition sportive, qu'il pratiqua dès son plus jeune âge, remportant, année après année, le cross de l'école primaire avant de devenir le champion de 400 mètres que vous avez évoqué, monsieur le président. Mais cet homme politique d'une redoutable pugnacité était aussi un homme chaleureux et sensible. L'un n'allait pas sans l'autre, et la longévité de son parcours illustre la confiance qu'il aura su inspirer à ses électeurs, pour lesquels il éprouvait un attachement sincère et réel. Il savait se montrer à l'écoute de chacun, avec une curiosité inépuisable et une profonde empathie. Après ses premiers pas dans l'enseignement à Ambarès, il fut élu conseiller municipal SFIO en 1965, à l'âge de 28 ans, puis succéda à René Cassagne en qualité de suppléant, devenant à 32 ans le plus jeune député de France, du département le plus grand de France En 1967, il devient président du conseil général, fonction qu'il exercera, à l'exception d'une période de trois ans, entre 1985 et 1988, jusqu'en 2015. Précurseur de la décentralisation, il crée en 1977 un fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, qui constituera un instrument d'aménagement précieux au service d'une exigence de justice et d'équité territoriales. Seul le Lot de Maurice Faure et la Nièvre de François Mitterrand s'étaient alors dotés d'un instrument comparable. Il manifesta ainsi précocement les qualités qui feront de lui le grand aménageur auquel les lois Defferre permettront de donner sa pleine mesure. « Pas de Gironde à deux vitesses », se plaisait-il à dire, et il mettra en place, au fil des années, les instruments permettant aux 535 communes de son territoire, qu'elles soient petites ou grandes, d'équipements structurants : places, salles polyvalentes, gymnases- tous ces lieux où se tissent les liens invisibles et indispensables qui font la cohésion sociale. En 2017, dans son discours d'ouverture de la séance publique, il portait un regard rétrospectif sur son action et disait avoir découvert, dans ses fonctions d'élu local, « l'importance déterminante du rôle des politiques d'aménagement et de solidarité mises en place par des institutions de proximité comme le conseil départemental À cette attention portée à l'équilibre territorial s'ajoutait un combat contre les inégalités. Philippe Madrelle s'investit tout particulièrement dans la politique de l'aide sociale à l'enfance, qui constitua l'un des axes de ses mandats de président de département et fut sa fierté, lui qui avait débuté sa carrière en tant qu'enseignant. Son territoire, il en avait une intime connaissance, connaissance des lieux, du patrimoine- du plus grandiose au plus modeste -, des élus aussi. Hervé Gillé, qui lui succède, a confié à la presse ses souvenirs de la campagne électorale de 2014, et son admiration de voir Philippe Madrelle appeler par leurs nom et prénom tous les maires et les adjoints rencontrés à cette occasion. Évoquant son souvenir, votre collègue Françoise Cartron a pu déclarer facétieusement : « Pas besoin de GPS avec Philippe Madrelle : il connaît toutes les routes de Gironde ! C'est fort de cet enracinement local que Philippe Madrelle deviendra député, puis sénateur. Après avoir siégé à l'Assemblée nationale de 1968 à 1980, il entra au Sénat et fut réélu à cinq reprises. Il y siégera près de trente-neuf ans. Ardent

Philippe Madrelle avait une longue expérience, mais ne se laissait pas entraîner à la facilité d'une nostalgie stérile. Il constatait les modifications profondes d'exercice du mandat parlementaire, en particulier, et des mandats politiques, en général. Il appelait de ses voeux l'approfondissement du travail des assemblées, tout en souhaitant que le Sénat puisse continuer à relayer les préoccupations de toutes les collectivités territoriales. Ce fut un homme qui suscita des vocations et forma des générations de jeunes élus talentueux et dévoués. Pour son territoire, pour la République, il eut la générosité de se projeter au-delà de lui-même. Il était conscient de la défiance manifestée par nos concitoyens envers nos institutions et ceux qui les incarnent, et appelait à la vigilance face à une lassitude des élus. Le projet de loi que le Sénat s'apprête à examiner lui aurait sans doute donné l'occasion de débattre avec le Gouvernement des moyens de conforter ces hommes et ces femmes politiques sans lesquels la démocratie ne peut fonctionner. Philippe Madrelle aura incarné une certaine génération d'hommes politiques, pour lesquels l'engagement était celui d'une vie. Fidèle à ses électeurs, fidèle à son parti, fidèle à son territoire, inlassable bâtisseur, il laisse un vide béant pour ses proches, pour son épouse, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs,

signe d'hommage à Philippe Madrelle, je vous propose maintenant d'avoir une pensée pour les quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, morts en service jeudi dernier et auxquels la Nation a rendu hommage ce matin.

Mes chers collègues, je vous indique que le Sénat sera appelé à se prononcer le jeudi 10 octobre, à dix heures trente, sur les conclusions de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable relatives à la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête afin d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen.

la parole sera accordée pour explication de vote à un représentant de chaque groupe pour une durée de deux minutes trente. Il n'y a pas d'observation ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, État et collectivités ont la République en partage. Les élus locaux, au premier rang desquels les maires, sont au plus près des citoyens, de leurs demandes, encouragements ou récriminations. Dans tous mes déplacements, je constate la volonté inébranlable de femmes et d'hommes portés par la fierté d'agir au quotidien pour leurs habitants. Ils conduisent leur mandat avec un engagement sans limite. Lors des consultations menées dans le cadre du grand débat national, les maires ont pu témoigner de cet engagement. Ils ont également confié leurs attentes et leurs aspirations. Ces attentes, je les comprends au regard de la complexité de la tâche à accomplir et de leur farouche volonté d'apporter à nos concitoyens les meilleures réponses à leurs problèmes du quotidien.

D'une part, il redonne des libertés locales, afin que les élus retrouvent des capacités d'action et que les décisions se rapprochent du terrain, en proposant une meilleure articulation entre communes et intercommunalités. D'autre part, il lève certains freins à l'engagement et au réengagement des élus locaux dans la perspective des prochaines élections municipales. Les propositions de ce texte sont résolument pragmatiques : elles visent à donner plus de souplesse et à remettre de la proximité dans l'exercice des politiques publiques. Ces actions sont très attendues au sein des territoires. Elles s'inscrivent dans la droite ligne de la mission que je mène à la tête de mon ministère : relever le défi de la cohésion des territoires. cette fin, nous avons renouvelé notre cadre d'action publique. Nous partons des besoins, des modes de vie locaux, pour proposer un accompagnement sur mesure des projets de territoire à travers les programmes d'appui. Nous travaillons en partenariat avec les collectivités territoriales pour revitaliser les centres-villes, promouvoir le retour de l'industrie dans nos campagnes, conforter le lien social et l'emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou encore assurer le déploiement du service public. De manière générale, nous voulons que chacun de nos concitoyens dispose des mêmes chances et des mêmes possibilités, quel que soit l'endroit où il habite. L'État devient facilitateur, accompagnateur des élus locaux, au lieu C'est ainsi que nous avons conçu l'agenda rural, que le Premier ministre et moi-même avons présenté au congrès des maires ruraux, le 20 septembre dernier à Eppe-Sauvage, dans le département du Nord. D'ailleurs, nombre de mesures inscrites dans le projet de loi que nous vous présentons aujourd'hui sont la traduction de mesures proposées dans cet agenda rural. C'est cette même philosophie qui guide les travaux préalables au prochain acte de décentralisation et de différenciation ; ce nouveau texte, appelé désormais « 3D »- décentraliser, différencier, déconcentrer -, vise plus largement à incarner les nouvelles relations entre l'État et les collectivités. Il permettra de développer une boîte à outils pour adapter notre action commune aux réalités locales. Il sera le réceptacle pour envisager de potentiels transferts de compétences entre l'État et les collectivités ou entre les collectivités elles-mêmes. Il sera également le réceptacle des mesures qui permettront, demain, d'assouplir la procédure d'expérimentation. Mesdames, messieurs les sénateurs,

La cohésion des territoires, objectif qui nous réunit, c'est le pari d'une France conquérante, parce qu'elle est attractive. Nous ne relèverons ce pari qu'en faisant alliance avec les collectivités territoriales, qui ont fait la démonstration de leur pleine maturité. Je n'en doute pas : le Sénat, dans sa grande sagesse, mettra tout en oeuvre pour renforcer ces libertés et responsabilités locales, comme il l'a encore signifié récemment. Ces enjeux sont tellement importants pour l'avenir de nos territoires qu'il nous faut y travailler collectivement, et de façon constructive ! La parole

Monsieur le président du Sénat, il y a maintenant quelques mois, je m'étais engagé auprès de vous à changer de méthodologie dans la construction du présent texte. Ainsi, nous avons mené des consultations directes avec les associations d'élus- nous en avons désormais l'habitude

en la matière dans notre pays, mais je crois que nous avançons et je tiens à m'en réjouir. La question de la formation est évidemment importante. Aujourd'hui, un élu départemental, régional, d'une grande métropole ou d'une grande ville,

dans leur commune : ils sont non seulement patrons de leurs collectivités territoriales, mais ils sont aussi officiers de police judiciaire, agents de l'État dotés de pouvoirs de police depuis maintenant plus de deux siècles. C'est un héritage de la Révolution française.

Comme vous le savez, quand j'étais maire de Vernon et président du conseil départemental de l'Eure, je m'étais opposé farouchement à ce texte. À juste raison ! Je resterai constant dans cette opposition. Ces trois

de montrer que, sur ces questions, nous savons parfois faire front commun. Ce qui est en jeu, c'est avant tout la démocratie locale et la vitalité de cette France communale. N'entendez pas dans mes propos une opposition entre l'intercommunalité d'un côté et la commune de l'autre ; pour nous, les choses sont claires : la commune, c'est la porte d'entrée de l'intercommunalité, l'échelon de base de la démocratie, le lieu

règne un esprit de coopération, de mutualisation et de projets. Ce bloc intercommunal est avant tout un couple, qui, avec le temps, devient indissociable, mais qui n'oublie jamais

il n'est pas question, aujourd'hui ou demain, que les membres des intercommunalités soient élus au suffrage universel direct. Nous avons fait la preuve de ce pragmatisme lors de l'examen de nombreuses dispositions

Mirabeau déclarait à l'Assemblée nationale qu'il fallait rapprocher l'administration des hommes et des choses ; en 2019, soit 230 ans plus tard, le mouvement des « gilets jaunes » et le grand débat national expriment, à leur manière, la même vérité. Mirabeau se serait-il donc fracassé sur l'atavisme jacobin de la quête du Graal d'un idéal égalitaire uniformisant ? Pour parodier Georges Brassens, « le temps ne fait rien à l'affaire » » ! Qu'avons-nous donc fait de la valeur unique et si précieuse de l'engagement des 600 000 élus locaux, ce long cortège de sentinelles de la République, et de ses valeurs ? Désenchantés, fatigués de réorganisations à marche forcée et de baisses des dotations, trop de maires réclament un cessez-le-feu en matière de big-bang territorial ; en même temps, tenus d'inventer des possibles pour leurs concitoyens et leur territoire, ils nous demandent d'effacer les irritants et de desserrer l'étau. Telle est votre volonté, monsieur le ministre, et je la salue d'autant plus sincèrement que le Sénat a quelque peu inspiré votre projet de loi. C'est avec cette même volonté de redonner aux élus une véritable capacité à agir, de retisser, au sein du bloc communal, des relations apaisées et positives,

est celui qui porte la responsabilité et qui en rend compte, celui qui est « à portée d'engueulade », comme aime à dire notre président. Le pacte de gouvernance, la conférence des maires, l'association des élus municipaux à la vie de l'intercommunalité sont de bonnes mesures, que nous saluons. Un second axe vise à donner à chaque territoire la possibilité de choisir le niveau le plus pertinent de l'action publique en sortant de cette rigidité normative parfois bloquante. N'est-ce pas là, monsieur le ministre, l'origine et la raison de votre projet de loi ?

que son territoire est trop vaste ou trop hétérogène ou que sa ville-centre est trop faible pour entraîner ses territoires ? L'intercommunalité a une vocation

Aussi le Sénat propose-t-il davantage de souplesse et d'agilité en supprimant la catégorie des compétences optionnelles, en ouvrant la voie à des transferts à la carte de compétences facultatives aux EPCI, en permettant d'inscrire dans la loi la procédure de restitution de compétences d'un EPCI à fiscalité propre. d'assouplir, de faciliter et de différencier pour permettre d'agir. Madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, lors du grand débat, le Président de la République a déclaré : « Il ne doit pas y avoir Il ne doit pas y avoir de tabou. » Il ne saurait donc y avoir de pré carré dogmatique intouchable ! Il y a juste, pour nous tous, une urgente et ardente obligation d'efficience de l'action publique dès lors que la République veut reconquérir le coeur de ses concitoyens. Votre texte est ambitieux, monsieur le ministre, vous entendez redonner confiance et envie aux élus locaux. Ici, dans cette chambre des territoires, en pensée avec le maire de Signes et avec tous les élus locaux, cette armée des faiseurs de la République du quotidien, nous vous disons, comme Mirabeau et sous le regard de Portalis, que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Alors, madame la ministre, monsieur le ministre, faites encore un effort pour nous rejoindre un pont plus loin : celui de la libre administration et de la responsabilité, celui de la confiance dans la République des territoires qui font la France ! La parole

en qualité de président de la délégation aux collectivités territoriales. Je mesure le caractère exceptionnel de cette prise de parole, que je prends comme une reconnaissance du travail de notre délégation, l'un des traits est l'investissement dans une coconstruction souvent fructueuse avec l'exécutif. Je veux saluer ici l'esprit de dialogue des ministres Jacqueline Gourault puis Sébastien Lecornu, avec lesquels nous avons travaillé très en amont du projet de loi. dès la finalisation du rapport de la délégation que nous avons présenté, en présence du président Larcher, en juillet 2018, des contacts ont eu lieu aux niveaux politique et administratif afin d'identifier très concrètement les pistes de mise en oeuvre. Nous avons pu mener ce travail préparatoire parce que

conduise une réflexion sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Cette démarche s'est faite en dialogue avec le Gouvernement, certes, mais aussi, et d'abord, avec les élus locaux. Nous avons fondé nos recommandations sur une longue série d'auditions, sur l'échange étroit et constant avec les associations d'élus, mais aussi, à la base, sur une consultation nationale des élus locaux de France, qui a reçu plus de 17 000 réponses. Du jamais vu a eu des effets concrets rapides pour les élus locaux, puisqu'un certain nombre de mesures réglementaires, avant même les projets de loi, ont mis en oeuvre, chemin faisant, sans tarder,

et, maintenant, un formulaire spécifique d'affiliation des élus locaux au régime général de sécurité sociale a été mis en place. De même, la prise en charge des frais d'hébergement des élus locaux, dans le cadre de leurs fonctions, a été améliorée. Ces avancées sont certes insuffisantes, mais elles remédient

nous avons engagé une mission pour mieux associer les élus municipaux à la gouvernance des intercommunalités. Sous une forme ou une autre, nous en trouvons l'écho dans ce texte dans

éviter d'aller trop loin vers de nouvelles obligations normatives au risque de rigidifier le travail des élus. Il en faut, mais pas trop ! Autant dire que, sur ces points, l'esprit du texte ne nous semble pas opposé à nos propres recommandations. C'est la raison pour laquelle nos amendements s'inscrivent dans sa dynamique. Je relève toutefois une exception, concernant la réécriture de l'article sur les modalités de fixation du taux maximal d'indemnisation des maires. Compte tenu des effets que ne manquerait pas d'avoir la mise en oeuvre de ces modalités, qui pèserait avant tout sur les plus modestes des élus locaux, ceux des petites communes, je ne peux que m'associer à la volonté de la commission d'infléchir la rédaction du projet de loi sur ce point. Je termine en saluant de nouveau le travail accompli par les collègues de notre délégation, toutes sensibilités confondues, en bonne intelligence avec les ministres et avec la commission des lois et je forme le voeu que cette convergence au service des élus locaux demeure à toutes les étapes du processus.

Dans le dossier de presse de ce projet de loi Engagement et proximité, vous écrivez : « Ce texte comporte des mesures concrètes, qui repartent de la vie quotidienne des élus, pour leur donner des marges de décision sur le terrain [ ...] et pour lever les freins à l'engagement ou au réengagement [ Objectif : clarifier le cadre d'exercice de leurs mandats alors que se multiplient les témoignages de maires qui ne veulent pas se représenter et qu'attirer de nouvelles personnes à l'engagement devient nécessaire.

que partagés. Néanmoins, le contexte est tout à fait particulier : une défiance s'est installée entre votre majorité et les territoires, qui s'est encore manifestée lors du congrès des régions à Bordeaux. Sachez que ce désamour est toujours d'actualité Dans une enquête commandée par notre groupe et réalisée en coopération avec le Cevipof, 27 % des maires interrogés font confiance au Gouvernement pour la mise en oeuvre des réformes locales, soit moins d'un tiers d'entre eux. état de cause, la première chose à faire est de vous féliciter de votre capacité d'adaptation puisque, en moins d'un an, nous sommes passés du hashtag #BalanceTonMaire au hashtag #CajoleTonÉlu ! #CajoleTonÉlu ! Si l'on était moqueur, ce dont vous ne pouvez me soupçonner, on ne pourrait que souligner l'heureux calendrier de ce projet de loi, qui, par le plus grand des hasards et parce qu'il est évidemment très utile, doit absolument être voté avant les élections municipales. Chacun sait ici que cette coïncidence est purement fortuite et que les propositions qui nous sont faites témoignent avant tout d'un intérêt sincère ... Quoique récent ! ... pour les maires et les élus locaux, intérêt que le Gouvernement tentera sans doute de prolonger jusqu'en septembre 2020. Sûrement ... Mais cela n'est que conjecture de ma part.

lèvres. Un texte parle aussi par ses manques ; nous y reviendrons. Abordons d'abord le couple communes-communauté. Vous présentez parfois l'intercommunalité comme une entrave

A-t-elle suscité parfois un sentiment de dépossession ? La réponse est oui ! Je suis un militant de l'intercommunalité, mais je constate qu'à certains endroits les élus peuvent se sentir perdus dans des grands ensembles. Faut-il alors corriger les périmètres « XXL » qui sont dysfonctionnels ? La réponse est encore oui, monsieur le ministre ! Il est toujours important de corriger et d'évaluer les effets d'un texte, en particulier ses effets pervers. Mais à l'inverse, faut-il se contenter d'une réponse qui peut s'assimiler à une remise en cause, alors qu'il faut avant tout permettre aux spécificités territoriales de s'exprimer ? La réponse est non ! Votre texte veut faire du « cousu main », mais il ne prend pas les mesures À ce sujet, vous avez vous-même reconnu, lors de votre audition au Sénat, qu'il était difficile de savoir combien d'intercommunalités allaient être concernées possiblement par les scissions. Après les irritants, vous vous prenez le risque de provoquer de nouvelles allergies. Il est plus important de travailler à la démocratisation des intercommunalités qu'à leur remise en cause. Faut-il prendre le risque de scission à un moment où les édifices se stabilisent ? Je ne le crois pas.

Je remarque juste qu'avant ce texte certains EPCI n'étaient pas en situation de mettre en place des politiques structurantes. C'est d'ailleurs probablement pour ce motif qu'une grande partie de cette assemblée- y compris à droite, bien que les intéressés aient tendance à l'oublier de manière fort opportune -, a voté le texte de la loi NOTRe. Vous l'aurez compris, si nous pouvons réfléchir à certains assouplissements correctifs, nous serons opposés à la remise en cause du couple communes-communauté. Comme le disait Pierre Mauroy, l'intercommunalité permet d'assurer un avenir à la commune. C'est bien aussi la solitude qui tue les petites communes.

dans le projet de loi de finances à remettre en cause les moyens dont ils disposent. Vous me direz qu'il faut attendre de nouveaux textes, notamment le « 3D ». Je ne suis pas sûr que les effets spéciaux suffiront à combler les élus locaux. Bien entendu, s'agissant des dotations financières, vous me renverrez à la diminution des dotations du précédent quinquennat. Oui ! On s'en Je vous rappellerai qu'elles ont été nécessaires essentiellement en raison des comptes publics, enfin, de ceux que nous avons trouvés en arrivant au pouvoir en 2012.

le texte initial, la logique indemnitaire que vous proposiez plaçait les élus devant un choix qu'ils ne pouvaient pas faire par manque de moyens. Il s'avère que le statut des élus, qui devait être le pilier de ce texte, n'en est plus qu'un élément, et c'est regrettable.

S'agissant enfin de la parité, vous évitez courageusement et avec détermination le sujet, bien aidé en cela par une droite qui a toujours eu du mal à supporter la fin du patriarcat en politique, et qui, à préfère payer 1,8 million d'euros plutôt que d'avoir plus de femmes élues. Mais la démocratie est aussi attaquée quand le texte rend facultatifs les conseils de développement. À un moment où on demande plus de participation, vous enlevez l'un des rares outils qui permet justement que s'exprime la diversité sociale. Pour conclure, monsieur le ministre, ce texte est-il mauvais ? Non, ? Non, mais il n'est pas en phase avec les objectifs que vous avez vous-même affichés. À vrai dire je suis très sévère, parce que

reste que, malgré ce jugement en demi-teinte, ce texte a le mérite de nous permettre de discuter tous ensemble de ces sujets. Certaines mesures seront utiles : je pense au pacte de gouvernance, à l'amélioration des prises en charge des frais de déplacement, éventuellement au vote des élus

tout en faisant en sorte de proposer d'autres améliorations parce que, encore une fois, nous aurions souhaité que l'ambition initiale soit respectée. Nous tenterons donc, avec les amendements du groupe socialiste et républicain, de faire progresser encore ce texte. La parole

en France, le maire est la pierre angulaire de notre culture républicaine, la clé de voûte de notre pacte social, le visage familier de notre quotidien. Il est l'élu préféré des Français. Mais malheureusement, depuis 2015 et le vote de la loi NOTRe, nos élus locaux se sentent dépossédés de leurs compétences. Que ce soit au profit des plus grands ensembles ou du fait de complexités administratives, le premier édile a vu son champ d'action se réduire alors que les attentes des citoyens à l'égard de son action municipale se font de plus en plus exigeantes. Les tensions exercées autour des budgets municipaux sont également sources d'inquiétudes. Malgré la prévision d'allocations compensatrices par le Gouvernement, l'avenir reste préoccupant pour nos maires baisse de dotation globale de fonctionnement, suppression des contrats aidés, incertitudes quant à la suppression de la taxe d'habitation et quant à l'équilibre du dispositif compensatoire, non-application de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévue dans le projet de loi de finances pour 2020 ... Comment en vouloir à nos maires d'être aussi interrogatifs ? Comment ne pas comprendre leur anxiété face à l'impossible équation de « faire mieux avec moins » ? Face à ces multiples défis, je ne peux donc que saluer l'initiative du Gouvernement de présenter un projet de loi visant à revaloriser la fonction de maire et son rôle au sein du modèle communautaire, à faciliter l'exercice de son mandat, notamment en étendant son pouvoir de police, et à susciter de nouvelles vocations pour un engagement local. Vous dire que ce texte était attendu, tant ici au Sénat, grand défenseur des collectivités territoriales, qu'au coeur de nos territoires, serait un euphémisme. Je regrette néanmoins qu'il manque de souffle pour l'avenir de notre modèle communal. J'espère donc que le Gouvernement sera sensible aux propositions formulées par le RDSE tout au long des débats pour remettre les maires au coeur de l'action, et la mairie, non pas au coeur du village-elle y est déjà-, mais au coeur de la République. Concernant la place du maire au sein du modèle intercommunal, ce texte de loi généralise des pratiques qui sont en fait déjà instaurées dans une grande majorité d'intercommunalités. Pour aller plus loin dans le pacte de gouvernance, le RDSE a souhaité introduire des amendements permettant d'y aborder certains sujets cruciaux, comme le schéma de mutualisation des services et le renforcement des solidarités financières. Nous avons proposé, dès le travail en commission, d'inclure le partage de documents essentiels aux fins de favoriser une bonne circulation de l'information au sein de tout EPCI pour l'ensemble des conseillers municipaux, ces exemplaires devant pouvoir être consultables en mairie, faute parfois d'accès informatique ou de réseau. Dans la version initiale du texte, le Gouvernement n'a pas souhaité aborder la question de la répartition des compétences. Malgré les frustrations générées par la loi NOTRe au sein de nos mairies, malgré l'objectif partagé de « conforter chaque maire dans son intercommunalité », seules les possibilités d'adaptation ou d'assouplissement sous contrôle de l'EPCI sont proposées. Il me paraît donc important de souligner le travail ambitieux mené par la commission des lois, l'initiative courageuse de ses rapporteurs, pour permettre un transfert de compétences à la carte. Le texte du Sénat supprime également le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement dans les communautés de communes et les agglomérations, ce que prônait le RDSE. C'est dans ce même esprit que j'ai souhaité déposer un amendement visant à conditionner l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal à un transfert volontaire et explicite de cette compétence « PLU » par la commune vers l'EPCI. Concernant le pouvoir de police du maire, le RDSE a tenu à vous soumettre des propositions concrètes. Ainsi, pour les débits de boissons, l'amendement déposé complète votre dispositif de fermeture en prévoyant que le maire puisse émettre formellement un avis simple et consultatif sur le dossier de demande d'ouverture des débits de boissons sur sa commune. Pour le défrichement, nous proposons aussi d'introduire un mécanisme d'information du maire. S'agissant de la gestion des épaves de voitures, la proposition du rapporteur d'une astreinte pesant sur le propriétaire est évidemment la bienvenue, mais, lorsque le propriétaire est inconnu, les frais restent à la charge de la commune. C'est pourquoi il est crucial de donner à la DGFiP un accès direct au système d'immatriculation des véhicules, le SIV, lui permettant d'identifier rapidement le dernier propriétaire de la carte grise, allégeant ainsi la procédure de recouvrement au nom des communes. Concernant la simplification du droit applicable aux élus, je tenais à vous remercier à cette tribune, monsieur le ministre, pour votre encouragement répété en faveur de ma proposition de loi visant au développement des médiateurs territoriaux dans nos collectivités. Intégré en commission à votre projet de loi, ce socle de médiation permettra, j'en suis persuadée, de faire prospérer un mode de règlement à l'amiable de conflits susceptible de faciliter ou de réinstaurer le dialogue entre les collectivités et leurs habitants. d'un outil de proximité, à l'image des élus locaux, au service du bien-vivre ensemble. Étant convaincue des bienfaits de la médiation, vous ne serez pas étonné de me voir porter également des amendements de défense et de promotion de nos conseils de développement. En conclusion, après cette scène 1, acte II des relations entre les collectivités territoriales, nous attendons avec impatience l'examen futur des textes annoncés par le Gouvernement sur la décentralisation et la différenciation, ainsi que sur la sécurité locale. Dans cette perspective, si notre groupe souhaite que le présent projet de loi Engagement et proximité soit une première pierre pour des textes plus refondateurs, il conditionnera son vote à l'adoption des amendements précités et au maintien des avancées introduites par la commission des lois. La parole est à M.

Nos démocraties connaissent depuis plus de vingt ans des transformations d'ampleur. Elles touchent aux clivages politiques, aux systèmes partisans, aux affiliations des électeurs et même à l'attachement aux libertés publiques. Tout semble bouger, dans une accélération du temps qui donne le sentiment d'une grande incertitude quant à la marche du monde, et favorise une forme de populisme par nature liberticide. L'horizon de l'idéal démocratique s'éloigne. Plus de 36 % des Français estiment qu'un autre système pourrait être aussi bon que celui de la démocratie. Les plus jeunes sont particulièrement favorables à une alternative à la démocratie. Nos concitoyens consentent à se départir des libertés publiques parce qu'ils sont inquiets, sans doute, face aux mutations climatiques, économiques, mais plus profondément, parce qu'ils se pensent moins comme citoyens que comme individus, prêts à ce que la liberté de tous s'efface pour peu que la leur soit garantie sous une forme de droit à jouir d'objets variés, de temps de loisirs, d'informations digestes. Pierre Rosanvallon appelle cela « l'individualisme de singularité ». Si la démocratie représentative est interrogée, je crois profondément en la démocratie territoriale, au plus près des besoins et des aspirations populaires, comme un moyen pertinent de convaincre nos compatriotes de se penser et d'agir en citoyens, comme un gage et un facteur de cohésion. Je voudrais remercier le Gouvernement de mettre la démocratie territoriale à l'honneur dans ce texte Engagement et proximité. Dans le droit-fil de cette réflexion, les élus locaux sont et seront plus encore le rempart face à ce mouvement indicible que j'évoquais. Ils renouent et renoueront avec le collectif face à l'individu. Nous avons plus que jamais besoin d'eux. Après avoir mis un terme à la baisse des dotations, stabilisé les moyens d'agir et stoppé les évolutions institutionnelles, le Gouvernement a souhaité les conforter dans leur rôle, consolider leur statut, clarifier leur environnement institutionnel. Ce texte comporte des mesures concrètes pour redonner aux élus, en particulier aux maires, la capacité d'agir plus librement, plus efficacement, plus simplement au quotidien meilleure gouvernance et information dans les intercommunalités, clarification des compétences dans le couple communes-intercommunalité, renforcement des pouvoirs de police du maire. Il comporte également des mesures pour lever les freins à l'engagement ou au réengagement : il s'agit des sujets d'indemnités, de formation, de prise en charge des frais de garde ou de protection fonctionnelle. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui procède en grande partie des travaux issus de notre assemblée, que ce soient des propositions de loi de nos collègues, de rapports issus de la commission des lois ou de rapports faits au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Je salue le Gouvernement qui nourrit sa réflexion des travaux du Parlement. Notre assemblée a été invitée à renforcer et à enrichir ce projet de loi, et la commission des lois a pu apporter des modifications substantielles. Les points C'est le cas par exemple pour le renforcement des pouvoirs de police du maire. Je me réjouis que notre amendement de suppression de l'article 42 de la loi NOTRe ait été adopté par la commission-il fallait qu'il le soit avant le 1 janvier puisque cet article article supprimait les indemnités d'un certain nombre d'élus dans les syndicats. Je me réjouis également que l'amendement visant à rehausser de 1 000 à 3 500 habitants le seuil de prise en charge par l'État des frais de garde

pour un amendement qui prévoyait un seuil plancher sur lequel le conseil municipal pouvait revenir. À titre illustratif, je suis un peu plus circonspect quant à l'adoption d'un amendement, qui me semble de circonstance, visant à autoriser les élus locaux à poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant leur arrêt maladie

trouver des dispositifs dont la décence n'est pas immédiatement caractérisée me semble un risque à éviter. En ce qui concerne la formation et l'aide à la reconversion des élus, la commission a accepté d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance tout en apportant des dispositions qui vont dans le bon sens, telles que la validation des acquis de l'expérience ou la possibilité pour le CNFPT de dispenser des formations aux élus. J'espère que nous évoquerons également le principe d'une formation socle qui pourrait être similaire à celle des agents publics, et pas seulement en matière de police judiciaire, mais aussi la possibilité d'être accompagné dans la perspective d'une fin de mandat pour une nouvelle carrière, voire une reconversion en valorisant les expériences acquises, ou encore les congés de formation. Enfin, s'agissant de la protection des élus, la commission a enrichi le texte initial tout en approuvant les mesures gouvernementales proposées. Je ne reviens pas dans le détail sur les dispositifs. Pour conclure, dirai que nous avons assisté jusqu'à maintenant à un travail collectif et constructif au sein de la commission des lois ; je ne doute pas que cet état d'esprit présidera à nos débats, dans l'intérêt des élus locaux dont nous sommes les représentants

quelques mots sur le département de l'Aube. Nous nous sommes intéressés à l'enseignement supérieur : tous les départements ne se sont pas intéressés à l'enseignement supérieur et, pour autant, si on ne l'avait pas fait, personne d'autre ne l'aurait fait à notre place. Nous nous sommes intéressés à des parcs d'activités départementaux

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues,

la poursuite des débats sur le texte des métropoles. Nous allons continuer à défendre l'idée que l'aménagement des territoires n'est pas la compétitivité entre eux, la suprématie de la métropole sur le reste. Au contraire, pour nous, l'urbain et le rural se complètent, l'État doit affirmer la solidarité entre les territoires tout en valorisant leurs atouts respectifs

que nous vivions dans notre pays précédemment. Nous avons donc le choix : nous pouvons mettre des pansements sur des plaies ouvertes et non refermées depuis plusieurs années, ou au contraire nous attaquer réellement à la problématique de l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, comme le titre de votre projet de loi nous y invite, Ce texte n'arrive pas au hasard. Il arrive en effet en milieu de quinquennat, après deux ans et demi de rapports que l'on peut qualifier de compliqués, parfois même conflictuels, entre le Président de la République, son gouvernement et les élus locaux. Il arrive également à un moment de crispation au sein de la société, après la crise des « gilets jaunes » et le grand débat qui a suivi, et qui, au vu des décisions prises et annoncées, Une fois de plus, et comme pour le grand débat, ce texte arrive à grands coups de communication. Pourtant, faut-il le rappeler, c'est un texte attendu par les élus et dont nous attendons tous des outils qui viennent en renfort de ces derniers. Le contexte doit être pris en compte, car nous avons connu ces derniers mois, voire ces dernières semaines, des épisodes d'agressions successives- je pense particulièrement à deux d'entre eux qui ont eu lieu dans mon département-et même un décès, avec la tragédie qui a touché la commune de Signes et son maire Jean-Mathieu Michel. Tous ces événements viennent donc inévitablement poser la question de la place de l'élu dans notre société, mais aussi des moyens que cette société lui donne dans l'exercice de son mandat. Ce point est très important, car il est un enjeu de la démocratie locale : il nous faut redonner du sens à l'action publique des élus envers les citoyens et les administrés. Le désengagement citoyen face à la perte d'engouement pour la participation politique n'est pas nouveau. L'abstentionnisme existait, mais il se renforce élection après élection. Les maires qui ne souhaitent pas renouveler leur mandat sont de plus en plus nombreux, d'où la nécessité de redonner du sens à cet engagement. Malgré les effets d'annonce, le texte initial qui devait être un grand projet de loi devient un simple ajustement technique où persiste à nos yeux un manque criant d'ambition. Le texte manque d'envergure : il répond certes à des problèmes particuliers, mais il ne répond pas globalement à la problématique de l'engagement des élus et de la population dans notre pays. Monsieur le ministre, vous l'avez vous-même rappelé dans vos propos pas de big-bang ni de grand soir. Mais d'ailleurs, en faudrait-il ? Sur ce sujet comme sur d'autres, l'histoire nous a démontré certainement qu'il ne le fallait pas. À la lecture précise de votre texte, votre texte, il n'y a que parcimonie, des avancées timides qui soulignent des problèmes criants sans les résoudre réellement et surtout dans la durée. Vous nous direz que tout ne relève pas de ce projet de loi et vous aurez raison. Vous nous direz d'ailleurs que de nombreux points évoqués seront traités plus tard, dans d'autres textes, que tel ou tel point relève du débat budgétaire. En bref, de vous-même, vous nous ferez comprendre que vous êtes loin de répondre aux attentes et d'apporter les solutions. Le texte aura alors suscité plus d'espoir que de résultats. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir qu'en politique susciter de l'espoir et ne pas y répondre est souvent dangereux. Alors d'ores et déjà, sachez que nous serons vigilants sur le projet de loi de finances, sur le futur projet de loi dit « 3D » que vous annoncez, madame la ministre, en espérant que nous ayons les bonnes lunettes pour pouvoir bien le lire, qui concernera la décentralisation, la différenciation et la déconcentration.

Si l'ambition affichée est réelle, il faut savoir dresser un bilan et en tirer les conséquences. Sans cela, il n'y aura ni rupture ni réorientation.

Rassurez-vous, mes chers collègues, l'heure n'est pas et ne sera pas aux règlements de compte ! Cela étant, faire de la politique, c'est un peu comme un récit de la mythologie grecque : il convient parfois de rappeler que ce sont toujours les choix des hommes

Ce texte peut être l'occasion de montrer ce que nous sommes capables de faire réellement pour les communes, les citoyens et les citoyennes. Voyez-vous, monsieur le ministre, il n'y aura pas de posture de notre part. Cela étant, dans votre intervention, vous avez cité

Et ce ne sont pas les maisons France services que vous annoncez qui viendront redonner du service public pour nos concitoyens, une présence de l'État pour accompagner les élus dans la réalisation de leurs projets.

collectivité. Comment s'engager quand il n'y a plus les moyens de porter des projets, le sentiment que tout se complexifie, que la proximité fait place aux grands EPCI et aux grandes régions ? Comment, dès lors, répondre aux besoins des populations ? La crise est là

Sachons revitaliser l'échelon communal et retisser le lien entre nos concitoyens et les élus. Telle doit être notre seule ligne directrice. Notre vote dépendra bien évidemment de nos débats. À nos yeux,

Ces diversités sont une chance : sachons incarner l'assemblée qui les fédère et qui ne les oppose pas. Évitons les clivages et les postures caricaturales entre campagne et ville.

Aussi, à cinq mois des élections municipales, le Gouvernement en nous soumettant ce projet de loi a l'ambition de replacer les maires au coeur de l'action publique locale et d'enrayer la crise des vocations.

de l'assainissement, de la voirie, du tourisme et du plan local d'urbanisme aux intercommunalités a donné aux maires et aux conseillers municipaux le sentiment d'être dépouillés et éloignés des décisions. Il est urgent de donner dès à présent aux élus la capacité d'agir, de décider librement et en responsabilité de la meilleure organisation pour leur territoire. En effet, le maire est l'interlocuteur naturel des administrés. Lorsqu'un habitant rencontre un problème, une difficulté, c'est au maire qu'il s'adresse spontanément, et non à l'intercommunalité.

Si le projet de loi que nous allons examiner vise à apporter des corrections à la loi NOTRe, afin d'en expurger un certain nombre d'« irritants », comme le disait M. le ministre, la commission des lois a amélioré très significativement ce texte, ce dont je me félicite.

le nombre de communes en France n'est pas un problème. Je crois même qu'il s'agit plutôt d'une chance. Je souhaite aborder plus particulièrement la question des compétences eau et assainissement. La loi NOTRe a prévu le transfert obligatoire de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1janvier 2020, malgré les réserves exprimées par le Sénat.

La loi du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a toutefois apporté quelques assouplissements bienvenus, sans être suffisants. Cette loi a permis aux communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas les compétences eau ou assainissement de s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles, si, avant le 1juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de cette communauté de communes, représentant au moins 20 % de la population, ont délibéré en ce sens. Je vous l'accorde, il s'agit d'une disposition extrêmement technique. Ce dispositif, qui institue une minorité de blocage, ne répond toutefois aux problèmes que de manière transitoire puisque, si ces conditions sont réunies, le transfert n'est repoussé que de six ans et prend effet au 1janvier 2026.

Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, et souligner la qualité de leur rapport. Particulièrement attentif aux préoccupations exprimées par les collectivités territoriales, notre groupe Les Indépendants demeure très attaché à une meilleure reconnaissance de la place centrale des maires et des élus,

Madame la présidente,

Sous Louis XIV, c'était « l'État, c'est moi ». Sous Napoléon, c'était « l'État d'abord ». Sous Clemenceau, c'était « l'État fait la guerre, je fais la guerre

au-delà des communes et des élus locaux, de se parler. On ne peut plus accepter cette parole qui vient d'en haut, quand elle peut être- c'est la démocratie ! -contestée et critiquée. En revanche, tous les citoyens

sinon le discrédit. Et les citoyens se sont sentis complètement écartés de la décision ! Tout à fait ! Aujourd'hui, il faut faire le travail inverse, non pas tout déconstruire

répondrai que ce pays tiendra d'autant plus que vous restituerez aux communes et aux 600 000 élus locaux leur capacité d'agir matérielle, financière, morale et intellectuelle. Retrouvons la démocratie

Jamais, depuis tant d'années, les communes n'avaient connu des changements aussi profonds dans une période aussi courte. Rappelons-en les principaux : la réforme territoriale et ses conséquences sur la réorganisation des territoires ; des nouveaux transferts de compétences que cette même réforme a entraînés ; la baisse des dotations de l'État et ses répercussions sur les budgets locaux ; enfin, la suppression progressive, partielle et bientôt presque totale de la taxe d'habitation, dont on ne sait toujours pas, de manière précise, par quoi et comment elle sera remplacée. Sans doute ces épisodes qui ont laissé un goût amer à nombre d'élus locaux ont-ils contribué à nourrir leur découragement, au point que l'on estime aujourd'hui que près d'un maire sur deux ne se représentera pas dans moins de six mois maintenant. Le projet de loi que nous nous apprêtons à examiner est-il de nature à réparer ce passé récent ? Pas vraiment. En effet, il ne revient pas sur les principaux griefs formulés à l'encontre des dernières réformes, qu'il s'agisse de la baisse des dotations ou des transferts de compétences imposés par la loi. est-il annonciateur d'une ère nouvelle dans laquelle les relations entre l'État et les communes seraient empreintes de plus de respect et de confiance mutuels ?

À l'évidence, oui, car toutes les propositions qu'il comporte vont dans la bonne direction. Celles-ci manquent quelque peu de souffle et d'envergure, mais elles apportent un petit plus pour les libertés locales, après les années de régression qu'ont imposées des lois venues de l'enfer. On sent comme un parfum de liberté dans ce texte, mais ce n'est qu'un parfum ! D'autres textes permettront au Gouvernement de montrer plus clairement ses véritables intentions. Je pense bien sûr au prochain projet de loi de finances qui, pour les collectivités, sera centré sur la question primordiale de la compensation de la suppression intégrale de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, mais aussi au nouvel acte de la décentralisation qui devrait intervenir au premier semestre de En attendant, ce projet de loi conforte le rôle du maire et de la commune. Il s'agit de l'une des réponses pour lutter contre la fracture territoriale dénoncée par les mouvements sociaux de ces derniers mois. Nous le savons, les Français aiment leur maire et leur commune plus que tous les autres responsables ou institutions politiques. Toutes les études le montrent, y compris celle qui a été réalisée par l'IFOP le mois dernier pour le compte de notre groupe,

Le conseil ou la conférence des maires n'est pas une nouveauté et donne satisfaction partout où il a été mis en place. Je crois à l'expertise, mais je crois plus encore à l'expérience. Voilà pourquoi je me réjouis que la commission des lois l'ait conforté.

dès lors qu'il en est d'accord, contribuera à un meilleur fonctionnement de la coopération intercommunale et, donc, à une plus grande efficacité de son action. faciliter la représentation des communes au sein des commissions de l'EPCI ou encore élargir la transmission des informations tenant aux réunions des conseils communautaires à l'ensemble des élus municipaux du territoire

Il est difficile d'expliquer aux maires que leur transfert a été imposé par la loi pour une plus grande efficacité, puis d'expliquer que cette efficacité passe par un retour à l'échelon communal. L'efficacité maximale eût donc été de ne rien faire Votre gouvernement n'est pas à l'origine de ce parcours, mais il avait la possibilité, l'année dernière, de sortir de cet imbroglio par le haut. Tel n'a pas été son choix et je le regrette. C'était avant, avant les mouvements sociaux qui l'ont amené à porter un regard nouveau sur les communes. Il n'est jamais trop tard, mais s'agissant de ces compétences, je pense que la commission des lois a adopté une position pertinente et cohérente, dans la droite ligne de ce qu'a toujours défendu le Sénat sur ce sujet. Je salue également la suppression de la révision automatique tous les six ans des schémas départementaux de coopération intercommunale. Le Président de la République l'a rappelé, les intercommunalités ne sont jamais que des constructions au service de la population. Elles doivent permettre aux communes de mieux répondre aux défis auxquels elles sont confrontées. La révision sexennale favorisait une logique de massification, notamment là où les préfets de département faisaient du zèle. Et il y en a eu ! Désormais, la carte intercommunale bénéficiera d'une certaine stabilité, ce qui donnera davantage de lisibilité aux EPCI et leur permettra de porter des projets à long terme. Enfin, ce projet de loi traite également du pouvoir de police des maires. Il propose d'ajouter à l'arsenal juridique existant quelques moyens nouveaux, dont la mise en oeuvre est aisée. L'efficacité devrait être au rendez-vous. Ce volet paraît mineur. Il l'est assurément pour les maires des grandes villes, mais il en va différemment des autres, qui ne bénéficient pas des mêmes services. Qu'il s'agisse des établissements recevant du public, de la tranquillité publique, de l'urbanisme opérationnel ou encore de comportements troublant la sécurité publique, tous ces domaines peuvent être sources de tensions qui empoisonnent le quotidien des élus. on ne les mesure pleinement que si l'on va les voir « avec les pieds », que si l'on prend le temps d'aller sur le terrain pour être à l'écoute. Précisément, l'écoute semble être la marque de fabrique de ce projet de loi, et c'est tant mieux

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, attendu de longue date, le projet de loi Engagement et proximité dont nous débattons aujourd'hui arrive à un moment choisi pour répondre aux attentes largement exprimées par les élus locaux et relayées depuis longtemps par le Sénat. Alors que les échéances de mars 2020 approchent, un maire sur deux hésite toujours à se représenter. Les raisons avancées sont toujours les mêmes : perte d'efficacité et d'utilité, absence de moyens et poids grandissant Cette situation est d'autant plus paradoxale que 67 % des Français font confiance à leur maire, bien plus qu'à leur député ou sénateur. Les causes de la baisse du moral des élus locaux sont connues : loi NOTRe, baisse des dotations durant le précédent quinquennat, multiplication et complexité des normes, désengagement des services de l'État. Et les inquiétudes pour l'avenir existent, notamment en raison du flou qui persiste autour de la réforme de la fiscalité locale. Formulées lors du grand débat, ces attentes ont été enfin entendues par le Gouvernement.

Je me félicite, comme l'a affirmé le Premier ministre au cours de sa déclaration de politique générale au Sénat le 13 juin dernier, que 80 % des dispositions de ce texte résultent des travaux du Sénat. C'est bien, mais peut mieux faire ! L'excellent travail de nos rapporteurs Mathieu Darnaud et Françoise Gatel contribue à enrichir le texte initial, afin de prendre en compte toute la réalité du vécu quotidien des maires et éviter que ce texte attendu ne rate sa cible. Conforter les maires dans leur rôle impose de redonner de la proximité à leur action et de favoriser leur engagement. La perte de proximité constitue un leitmotiv. Beaucoup de maires rencontrés affirment être trop souvent dépourvus face à des décisions intercommunales prises sans leur consentement, ou des mesures législatives ou réglementaires déconnectées de la réalité et appliquées uniformément par les préfets. L'application du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie en Seine-Maritime en est une parfaite illustration. Plus récemment, la faible information des maires lors de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen- je pense à ma collègue Catherine Morin-Desailly - a privé la chaîne de communication auprès des citoyens d'un maillon essentiel, relais de proximité nécessaire.

et de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, il tend à rééquilibrer les relations entre communes et EPCI pour que l'intercommunalité soit au service de la commune, et non l'inverse. Souhaitant aller plus loin, la commission des lois a renforcé la place de la commune, en autorisant le transfert de l'intercommunalité vers la commune de compétences ou de la gestion d'équipements de proximité. Cette nouvelle souplesse permettra d'adapter l'organisation des EPCI aux spécificités locales, de faire du sur-mesure et d'éviter le modèle unique. Si la proximité est essentielle pour redonner du sens à l'action municipale, elle ne peut suffire pour favoriser l'engagement des maires. L'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux est vitale pour encourager les vocations et favoriser l'engagement en politique, notamment des femmes. Seuls des femmes. Seuls 16 % des maires sont aujourd'hui des femmes ; on ne peut que le déplorer. La conciliation de la vie professionnelle, de la vie politique et de la vie familiale reste difficile. La prise en charge des frais de garde et de déplacements est une première avancée.

L'augmentation du plafond des indemnités réclamée par les élus doit rester supportable par les budgets communaux et acceptable par les administrés. C'est tout le sens des améliorations introduites par les rapporteurs. Enfin, la perte de ressources et de cotisations retraite liée à l'engagement politique et la gestion de la fin de mandat restent de véritables sujets de préoccupations pour les élus locaux, sur lesquels nous devons encore progresser

nous sommes à cinq mois des élections municipales et nous avons compris qu'il était temps, pour l'exécutif, de tenter de combler le fossé qu'il a creusé avec les élus locaux, l'éloignant des territoires. les décisions négatives se sont multipliées depuis le début du quinquennat, suscitant interrogations, inquiétude, défiance et, parfois, colère. Dès 2017, alors que le Président de la République affichait sa volonté de dialogue avec les élus locaux en instituant la conférence des territoires, le Gouvernement annonçait, sans concertation, l'annulation de plus de 300 millions d'euros de crédits d'investissement dédiés aux collectivités. C'était mal parti Suivaient la diminution drastique du nombre d'emplois aidés, amputant les politiques d'insertion, affaiblissant les associations et obligeant les communes à voler à leur secours, la baisse des APL, impactant le modèle économique des HLM et, par conséquent, les politiques d'urbanisme et de logement des maires et, enfin, la disparition de services publics locaux, celle des trésoreries en étant le dernier avatar. Puis- je vous passe des étapes -est venue l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation, qui fera l'objet non pas d'un dégrèvement, mais d'une compensation par transfert de fiscalité, rappelant la suppression, de triste mémoire, de la taxe professionnelle et ses conséquences sur les finances locales. Enfin, cerise sur le gâteau, le hashtag #BalanceTonMaire a démontré toute la considération du Gouvernement et de la majorité pour les 600 000 élus locaux qui, chaque jour, s'engagent au bénéfice de leurs concitoyens et de leur territoire. Il aura fallu la crise des « gilets jaunes » et l'appel à la rescousse des maires pour que le Président de la République découvre qu'ils étaient indispensables au lien social, à la cohésion territoriale et, tout simplement, à la République, dont ils sont bien souvent le rempart. C'est à cette occasion que M. Macron a découvert que nos collègues étaient en souffrance et qu'ils avaient le, à tel point que nombre d'entre eux n'envisageaient pas de se représenter et que l'on pouvait craindre une crise des vocations. Ce texte arrive, par un pur hasard de calendrier, juste avant les échéances municipales et sénatoriales de 2020, avec l'ambition affichée de répondre aux attentes des maires, de retisser du lien, de redonner confiance. Nous ne sommes pas dupes de la manoeuvre, mais, en responsabilité, nous sommes prêts à prendre tout ce qui améliorera la vie de ces élus, même si le projet de loi est loin de répondre à l'ambition affichée.

Enfin, ils veulent retrouver de la liberté d'action, sans contractualisation étouffante, sans tutelle suffocante des services préfectoraux, sans avalanche de normes nouvelles. ministre, monsieur le ministre, vous avez fait le choix de reprendre de nombreuses dispositions déjà votées par le Sénat, souvent à l'unanimité, qui, malheureusement, faute de relais au Gouvernement et au sein de la majorité de l'Assemblée nationale, n'avaient pas pu prospérer.

Plusieurs de nos propositions ont été reprises, essentiellement sur les droits des élus. Nous nous en félicitons. Nous présenterons, en séance, d'autres amendements, qui, nous l'espérons, pourront rassembler. concerne la consolidation de la place de la commune et du maire dans l'intercommunalité, nous invitons nos collègues à aller plus loin que nos rapporteurs, en rendant obligatoires le pacte de gouvernance et la conférence des maires, considérant que c'est dans les territoires où ils n'existent pas encore qu'ils seront les plus utiles et que, sans obligation, il y a peu de chances qu'ils y voient le jour. Nous veillerons, par ailleurs, à ce que les possibilités de scission d'EPCI soient bien réservées aux quelques cas d'intercommunalités « XXL » posant difficulté, en fixant des bornes quant à leur taille, à leur taille, et à ce que l'assouplissement de la répartition des compétences n'ouvre pas de remise en cause insidieuse de l'intercommunalité. Il ne faudrait pas que la suppression des compétences optionnelles

des conditions d'exercice des mandats locaux, nous nous félicitons que la commission ait retenu notre proposition selon laquelle seul le maire peut demander une indemnité inférieure au plafond. Nous aurions souhaité que les indemnités des maires et des adjoints puissent être augmentées de façon dégressive, au-delà de 3 500 habitants jusqu'à 100 000 habitants, au-dessous de laquelle l'indemnité du maire est inférieure au salaire médian français. Très bien ! De nombreuses autres dispositions vont dans le bon sens, bien qu'elles ne révolutionnent pas le quotidien des élus et que ce soit au final le budget communal qui devra, s'il en a les moyens,

des manques, notamment sur la parité, alors que ce texte devrait permettre de la faire progresser au sein des EPCI, qui ne comptent qu'un tiers de femmes et seulement 8,9 % de femmes présidentes.

alors que c'est une condition de l'engagement. Qu'en est-il de la validation des acquis de l'expérience ? Qu'en est-il de la reconversion professionnelle ? Sur ce plan, nous aurions souhaité que le texte prévoie le bénéfice de l'ancienneté des élus dans le cas d'une reprise d'activité, amplifie l'allocation différentielle de fin de mandat, soutienne la création d'entreprise, en faisant bénéficier l'élu de prêts en quasi-fonds propres. Nous aurions aussi voulu réformer le régime de retraite des élus, alors que celle-ci est, aujourd'hui, indigente. Ces sujets ne figurent pas dans le texte, et l'article 40 de la Constitution ne nous permet pas de les y intégrer. Nous regrettons que le Gouvernement n'en ait pas pris l'initiative. Madame la ministre, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, la question de l'engagement citoyen est primordiale. Ce texte va-t-il décider des élus sortants hésitants à se représenter ? Va-t-il susciter de nouvelles vocations ? Nous ne le croyons pas. Il ne règle en rien la question des moyens financiers. Il ne règle pas plus celle d'une liberté retrouvée

Bref, notre République s'appuie sur ces élus, qui offrent à notre pays un véritable équilibre, une paix dans un contexte pour le moins agité. Si l'on peut débattre de leur nombre au sein du conseil municipal quand on connaît la difficulté qu'ont certains candidats à constituer une équipe,

Le « statut de l'élu » est-il devenu un gros mot ? Avons-nous peur des citoyens ? Depuis des années, les élus locaux revendiquent un statut. Pour rappel, ce terme n'a rien de subversif ! Il s'agit uniquement d'un ensemble de textes qui règlent la situation d'une personne ou d'un groupe.

Les enjeux du statut de l'élu sont triples. Alors que plus de deux maires sur cinq sont des retraités, alors que seulement 16 % des maires sont des femmes, ces enjeux sont ceux de notre société : il s'agit de lutter contre les freins à l'engagement liés à l'activité professionnelle, à la parité et à la représentation de la société dans la vie publique.

Une quantification du temps qu'exige l'exercice d'un mandat municipal s'impose pour expliquer aux citoyens la nécessité de réformer les retraites et les indemnités des élus locaux. À cet égard, ce texte aurait dû associer les droits et les devoirs. Comment, dans un contexte social en crise, dans une défiance exacerbée des citoyens envers leurs gouvernants, imaginer des droits sans devoirs ? Alors que le « tous pourris » inonde les réseaux sociaux, les élus locaux font les frais de ce manque de confiance, mais également de l'absence de respect, qui s'amplifie.

92 % des participants à la consultation ont déjà subi des incivilités, des injures, des menaces ou des agressions physiques. Rédiger des textes de loi pour renforcer les moyens de contrainte, c'est bien. Expliquer, c'est essentiel, car la citoyenneté ne se décrète pas, pas plus C'est pourquoi nous devons collectivement oeuvrer pour reconquérir les Français. Nous devons collectivement débattre, expliquer, quels que soient nos mandats et quels que soient les publics. Pourquoi, par exemple, ne pas imposer à chaque élu de consacrer une demi-journée par mois à une rencontre avec les jeunes ? La citoyenneté se crée dès le plus jeune âge, et je peux vous dire, pour rencontrer les conseils municipaux de jeunes, mais également des élèves et des étudiants du CE2 jusqu'au master 2, qu'il y a une vraie appétence pour nos institutions.

J'ai réalisé une enquête dans mon département : 82 % des maires qui ont répondu y sont favorables. D'après ce même questionnaire, pour 74 % des maires, l'exigence accrue des citoyens représente le principal frein à l'engagement. C'est pourquoi il est fondamental de témoigner, d'informer sur le rôle majeur de nos élus et de soutenir encore et toujours cet extraordinaire maillage de notre pays. En ce sens, le groupe RDSE a déposé de nombreux amendements qui vont plus loin que le texte examiné, car, si le débat a le mérite d'être posé sur plusieurs sujets, certaines propositions sont perçues par les élus locaux comme des effets d'annonce ou de communication. Par exemple, quelle valeur aura la possibilité, pour un EPCI, de déléguer la compétence eau et assainissement aux communes qui le souhaitent, si cette délégation est soumise au vote de

loin. L'augmentation du pouvoir de police du maire est également une bonne intention. Toutefois, dans la réalité, certains pensent que cela les mettra encore plus en danger. Mais non ! Un accompagnement par les services d'État est donc nécessaire.

le projet de loi qu'il nous est donné d'examiner aujourd'hui marque une prise de conscience par le Gouvernement du rôle des élus locaux dans notre démocratie et de la nécessité de mieux les considérer. chez les élus, un sentiment latent de dépossession s'est installé. Successivement, ils ont dû affronter les baisses de dotations de l'État, qui ont affecté toutes les collectivités de manière indistincte et non concertée, puis la marche forcée vers les grandes intercommunalités et les grandes régions et, demain, la réforme de la fiscalité locale. Ce projet de loi entend ainsi valoriser et accompagner ceux qui s'engagent pour la démocratie et la collectivité, en améliorant les conditions d'exercice des mandats locaux. Dans le même esprit, il vise à étendre les libertés locales, à conforter le rôle du maire pour assurer un meilleur équilibre avec l'intercommunalité, à simplifier le quotidien des élus locaux et à mieux adapter certaines règles ou certains seuils aux réalités territoriales.

Il est primordial de faire de l'intercommunalité un véritable instrument au profit des maires. N'oublions pas que ce sont les communes qui font l'intercommunalité, et non l'intercommunalité qui fait les communes Je suis heureux également que ce projet de loi prévoie de lever des freins à l'engagement et au réengagement, pour attirer de nouvelles personnes à se présenter et pour ne pas décourager les élus locaux, alors que la menace de voir des listes incomplètes aux élections de 2020 se fait jour. toutefois qu'il faudrait aller plus loin. En effet, sur le terrain, les maires, notamment ceux des communes de moins de 1 000 habitants, réclament une diminution du nombre de conseillers municipaux, car ils rencontrent des difficultés à constituer des listes en vue des prochaines élections.

De plus, l'abaissement du seuil du scrutin proportionnel en contrepartie, en le fixant, par exemple, à 200 habitants, favoriserait la parité et la démocratie et réduirait l'iniquité qui existe actuellement pour le même scrutin. En effet, pour les communes de 1 000 habitants

au premier rang desquels les maires, qui sont toujours au plus près des citoyens, de leurs demandes, de leurs encouragements, mais aussi de leurs récriminations. Oui, le travail que mènent les élus au quotidien au service des habitants, au niveau communal comme au niveau intercommunal, doit être simplifié et soutenu. Oui, le bloc communal doit être valorisé et remis au coeur de notre démocratie. C'est une valeur essentielle de notre République ! Monsieur le ministre, mes chers collègues, réenchanter l'exercice de ce bel engagement qu'est le mandat local est à portée de main.

Rendre l'engagement citoyen attractif pour de nouveaux élus et répondre aux demandes des maires d'aujourd'hui : voilà l'urgence à laquelle ce texte doit répondre. Pour cette raison, le groupe Les Indépendants votera

parce qu'il traite de la difficile et nécessaire représentation locale de l'ensemble de nos concitoyens. Essentiel, parce qu'il touche le socle même de notre modèle démocratique. Essentiel, enfin, parce qu'il rappelle le rôle premier de notre chambre, tel qu'énoncé à l'article 24 de la Constitution française : celui d'assurer la représentation des territoires de la République. Assurer leur représentation, c'est accompagner les élus locaux dans l'exercice de leurs missions ainsi que dans la gestion de leur commune, dont ils connaissent mieux que quiconque les réalités, les exigences et les turpitudes du quotidien.

Malgré la volonté affichée de décentralisation, l'atavisme jacobin rattrape malheureusement trop souvent les 35 000 communes qui composent notre territoire. Le trouble est important pour les élus locaux, qui assurent avec beaucoup de dignité des fonctions parfois difficiles. Surtout, la nature et le rôle de l'élu s'en trouvent considérablement transformés. Ces dernières années, nous avons bien senti dans nos territoires une forme de découragement, qui a saisi de nombreux élus. Ce découragement est engendré par le décalage entre l'envie d'agir des élus et les trop nombreux obstacles auxquels ces derniers doivent faire face, se sentant souvent trop seuls face à la complexité de nos organisations institutionnelles et la diminution des moyens de nos collectivités territoriales. Les fonctions que nous occupons aujourd'hui au Sénat, celles que nous exercions hier dans nos communes, comme maires, adjoints au maire, conseillers municipaux, départementaux ou régionaux, nous ont placés quotidiennement au contact de la France des élus locaux, de l'engagement, du courage et de la prise de risque, celle des communes, grandes et petites, celle des petits bourgs, des communautés d'agglomération et des métropoles. C'est pourquoi nous mesurons, mieux que d'autres peut-être, le gâchis des énergies contenues dans nos territoires. cette position privilégiée, à cette tribune comme dans les allées des marchés, nous mesurons à quel point la volonté, l'abnégation et le sens du mouvement se heurtent à chaque instant aux forces du statu quo. Non, gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages n'est pas chose facile. Sur ce plan, les échanges constructifs entre le Gouvernement, quel qu'il soit, et le Sénat sont une école de réalisme : on n'administre pas un pays contre ses élus locaux. Oui, la condition de nos élus locaux se dégrade. De nombreux exemples nous l'ont malheureusement montré. D'abord, les efforts à fournir pour assurer une fonction dont l'indemnisation est faible au regard du temps consacré et des efforts consentis la délégation de compétences aux EPCI et la diminution des moyens mis à la disposition des communes nourrissent les tensions, les incompréhensions et, à terme, les divisions entre les élus et leurs administrés, dont les problématiques, aux facteurs éminemment locaux, trouvent rarement une réponse simple, concrète et efficace. La dégradation de la fonction d'élu doit être une préoccupation majeure pour notre assemblée, parce que nous sommes les représentants des élus, mais aussi et surtout parce qu'une remise en cause du rôle de l'élu local est une mise à mal de notre socle démocratique. L'élu local et la commune étaient au coeur des grandes avancées vers la décentralisation de notre pays. Les lois Defferre constituèrent des avancées considérables pour la démocratie. Les récentes tentatives de décentralisation sont, elles- il faut le reconnaître -, bien plus floues. En effet, la décentralisation a conduit à un enchevêtrement des compétences, qui obscurcit les réalités et dilue les responsabilités. Aujourd'hui, posons-nous les bonnes questions.

d'une confiance en la capacité de notre assemblée à se saisir de sujets aussi importants pour la démocratie locale. C'est dans cet esprit de confiance et de proximité que nous assumerons pleinement notre rôle.

Il apporte, au titre I, la nécessaire clarification du rôle des maires dans les EPCI, à travers la possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance ainsi qu'une conférence des maires.

C'est un point fondamental. L'exercice d'un mandat permet d'acquérir de nombreuses compétences. Celles-ci doivent être reconnues. Une élection ne peut plus être un frein ou une parenthèse dans une carrière professionnelle. À ce titre, les actions de réinsertion doivent faire partie des formations financées sur les budgets locaux, dans l'enveloppe de formation déjà prévue par le code général des collectivités territoriales. Il s'agit ainsi d'encourager la réinsertion des élus, et donc la fluidité de leur carrière professionnelle. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant le débat. En pratique, ces formations restent très peu mobilisées. Les élus locaux doivent être mieux accompagnés dans leur reconversion professionnelle, notamment par la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Il s'agit d'assurer la cohérence entre cet outil de formation et le DIF.

Ce texte se veut une réponse au mal-être des élus. Il ne réglera pas la question dans son intégralité : les problèmes sont si divers que la réponse ne peut être unique. Madame, monsieur les ministres, vous affirmez l'ambition de clarifier le rôle de l'élu dans un cadre qui a évolué et de concevoir l'élu local que nous voulons pour demain. Notre société ayant changé, les élus locaux, eux aussi, sont amenés à évoluer. Ils aspirent désormais à plus d'autonomie et de responsabilité, dans tous les domaines. Cela est encore plus vrai des nouvelles générations qui arrivent. Par plaisanterie, on a pu dire de la politique qu'elle était l'art d'empêcher les gens de s'occuper de leurs propres affaires. Il nous faut aujourd'hui faire tout le contraire. L'exigence pour les prochaines années, c'est la redistribution des pouvoirs. il n'y aura pas de partage des pouvoirs sans véritable décentralisation. Le mot reste cependant ambigu : il accrédite l'idée que les pouvoirs viennent d'en haut et que c'est le sommet de l'État qui décentralise « ses » pouvoirs au profit des collectivités territoriales. La décentralisation cache souvent une simple déconcentration déconcentration des pouvoirs. Il nous faudra remettre la décentralisation à l'endroit. Ce texte peut être une première pierre à l'édifice. Les échanges qui suivront doivent viser à présenter une analyse de la situation, à donner du sens à notre action et à montrer sur quoi peuvent déboucher les efforts de nos élus.

à celles, pas encore élues, qui se posent la question de leur présence sur une liste municipale. Simplifier la gestion de nos communes, élargir de nouveau le champ des possibles pour les élus, redonner du sens et de l'envie à l'engagement

Mes propositions visent à rendre hommage à nos maires, à nos élus locaux, afin de les valoriser et de susciter des vocations. Ils sont avant tout enracinés dans leurs territoires, dévoués à leurs concitoyens et passionnés par la vie publique. Donnons-leur la reconnaissance qu'ils méritent

Il est impératif de communiquer sur cet engagement au service du bien commun. Troisième constat, face aux grandes intercommunalités, nos élus se sentent exclus, privés de parole, et donc démotivés.

Nos maires se sentent déshabillés. Il est essentiel de redonner du pouvoir de décision à nos élus. Je salue à cet égard le travail de nos rapporteurs. Fidèle à l'esprit du Sénat et à sa connaissance du terrain, a supprimé le transfert obligatoire de la compétence en matière d'eau et d'assainissement- une aberration que nous n'avons de cesse de dénoncer. Le Gouvernement entendra-t-il raison à ce sujet ? Le cinquième constat concerne les indemnités et leur caractère dérisoire au regard des responsabilités des maires de nos petites communes, taillables et corvéables à merci

De nombreux élus locaux vivent, selon leurs propres mots, un « véritable malaise » et une « crise des vocations ». En effet, le poids des responsabilités et la complexité de leurs missions n'ont cessé de croître, alors que leur statut, notamment leur indemnisation, n'a pas évolué en parallèle. Ce projet de loi peut nous permettre d'y remédier, et je remercie les rapporteurs pour leur travail sur ce sujet. Garder les trois premières strates actuelles, telles qu'adoptées en commission, me paraît aussi nécessaire pour la cohérence et l'acceptation de la valorisation indemnitaire. Cette reconnaissance passe aussi par certains symboles, notamment quand d'autres élus locaux et nationaux en bénéficient déjà. Je pense ici à la cocarde tricolore, que nos maires ne peuvent rendre visible dans leur véhicule sous peine d'être verbalisés, comme le fut le plus ancien maire de mon département, après cinquante ans de mandat

La récente consultation sénatoriale auprès de nos édiles montre que ces faits divers sont une réalité trop répandue. Nos maires, pourtant officiers de police judiciaire, vivent mal le classement sans suite de plaintes et les procédures judiciaires sans fin, alors que la responsabilité pénale du maire est trop souvent engagée.

Mon septième constat est celui du manque de sécurité, qui entraîne une crise des vocations. Certes, être élu n'est pas un métier ; toutefois, pour susciter des vocations, il faut rendre la fonction plus respectée et attractive.

Il faut aussi faciliter la mise en disponibilité, pour l'exercice de leur mandat, aux élus salariés du privé, sur les mêmes bases que pour les agents de la fonction publique. La problématique est abordée dans le projet de loi, mais celui-ci renvoie à des ordonnances. Enfin, à propos de proximité, on ne peut que déplorer,

possible le cumul de mandats, de renforcer le lien unissant les territoires à leurs représentants nationaux. Madame, monsieur les ministres, mes chers collègues faisons en sorte que le texte qui sortira des travaux du Sénat soit à la hauteur des attentes de nos maires ! C'est l'intérêt général qui guide l'action de nos élus locaux leur engagement mérite une reconnaissance pleine ; cela est légitime et juste

C'est vous dire combien j'étais sinon impatiente, du moins curieuse, madame, monsieur les ministres, de découvrir le grand projet de loi annoncé par le Gouvernement et destiné -je cite l'exposé des motifs -« à lutter contre la fracture territoriale » et « à réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural » : rien de moins ! Personne n'est dupe de cette « opération séduction » lancée à quelques mois des élections municipales, et il faudra bien plus qu'un projet de loi pour renouer la confiance avec les maires et les élus locaux. Ainsi, il aura fallu la crise des « gilets jaunes » pour que l'exécutif se rende enfin compte des difficultés rencontrées au quotidien par les maires, expliquant pourquoi un maire sur deux déclare ne pas vouloir se représenter lors des élections municipales Oui, les communes sont le socle de la République, les maires sont les premiers agents de l'État sur le territoire : un État qui, sans les élus locaux, serait bien en peine de préserver la cohésion sociale. Aujourd'hui, pardon de le dire, ils sont bien mal payés en retour avec ce projet de loi. En effet, malgré les intentions affichées par le Gouvernement, le compte n'y est pas : rien sur les baisses de dotations de l'État, ni sur la suppression de la taxe d'habitation, qui bat en brèche l'autonomie financière des collectivités territoriales, pourtant inscrite dans la Constitution peu de choses sur les intercommunalités « XXL » et rien sur les super-régions qui éloignent le pouvoir du terrain et laissent les élus communaux seuls en première ligne ; service minimum sur l'assouplissement maintes fois annoncé de la loi NOTRe ; rien sur l'acte III de la décentralisation que réclament en vain les associations représentatives des communes, des départements et des régions ; surtout, rien sur ce qui constitue le vrai problème, qu'avec la réforme territoriale et la priorité donnée au couple intercommunalité-région, avec la marche forcée vers les grandes intercommunalités, la légitimité technique par la compétence est, peu à peu, en train de remplacer la légitimité politique par le suffrage. Place aux « technotables » ! Telle est la vérité du malaise des élus locaux, et pas seulement des maires. Vous dites vouloir donner plus de pouvoirs aux maires, mais ce n'est pas en les autorisant à fermer les débits de boissons à la place des préfets que vous rétablirez la confiance. surtout à soulager une fois de plus les services de l'État d'une tâche subalterne et à placer les maires dans des situations délicates. Donner des pouvoirs aux maires ? Mais pour faire quoi, et avec quels moyens ? Ce que nos collègues élus locaux réclament, c'est déjà de pouvoir disposer de moyens suffisants pour exercer leurs responsabilités actuelles. Commençons par là : ce serait déjà bien. C'est en tout cas que m'ont répondu les maires de la Haute-Savoie que j'ai pris soin de consulter sur la base de votre projet de loi et dont je me fais l'interprète aujourd'hui. Enfin, à quoi bon vouloir légiférer tout le temps et sur tout ? Je fais ici référence au projet de pacte de gouvernance et à la conférence territoriale des maires, qui se pratiquent déjà sous des formes diverses sur le terrain sans qu'il soit besoin de loi pour cela, tout simplement parce que la solidarité entre les territoires et la confiance entre les élus locaux ne décrètent pas, mais se vivent au quotidien. Le vécu quotidien des maires et de leurs adjoints- ne les oublions pas c'est souvent le choix de ne pas percevoir ses indemnités pour ne pas grever un budget communal déjà faible. À cet égard, le relèvement du plafond des indemnités que vous proposez et dont vous laissez la modulation à la discrétion des maires est une réponse insuffisante. Le vécu quotidien des maires et des adjoints, c'est la difficulté à concilier vie professionnelle, vie familiale et mandat électif, en particulier pour les femmes, nombreuses à être engagées dans la vie publique locale. Le vécu quotidien des maires et de leurs adjoints, c'est le maintien coûte que coûte d'un service de proximité et de qualité répondant aux besoins de leur population. Quand j'entends le Gouvernement annoncer la création de plusieurs milliers de maisons des services au public, tout en laissant leur fonctionnement futur à la charge des communes, je réponds qu'il existe déjà près de 35 000 maisons des services au public en France : cela s'appelle les mairies ! Le vécu des maires et des adjoints, c'est le temps qui manque pour se former et la difficulté à conserver une activité professionnelle régulière et, le cas échéant, à retrouver une activité ou à se reconvertir en fin de mandat.

Madame, monsieur les ministres, nous autres montagnards sommes des taiseux ; nous ne donnons pas notre confiance comme cela, nous jugeons aux actes. Comme se plaisait à le dire Churchill, « que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder Comme beaucoup de mes collègues, j'attendrai donc de voir quelle suite vous réserverez aux propositions du Sénat pour me prononcer. Il ne tient qu'au Gouvernement de faire en sorte que ce débat ne soit pas une occasion manquée. La parole

comme le soulignait fort justement le président de la Haute Assemblée, Gérard Larcher, « le temps est venu de recréer des ponts entre les collectivités territoriales et l'exécutif En effet, le lien de confiance entre les élus locaux et l'État a été fortement et durablement endommagé. Disons-le sans ambages, il ne tient plus qu'à un fil. Les dégâts occasionnés par le chamboule-tout des réformes territoriales bâclées, le des contraintes financières étranglant l'autonomie fiscale locale, les ravages causés par les mensonges de la Conférence nationale des territoires, l'ignominie du hashtag #BalanceTonMaire doivent être réparés maintenant ! En point d'orgue de cette vertigineuse dégradation, la grave crise dite des « gilets jaunes » est venue stopper net l'arrogance du « nouveau monde » et a plongé le pouvoir dans la crainte et la fébrilité. Après avoir fait un chèque sans provision de plus de 10 milliards d'euros pour acheter la paix sociale, le Président de la République s'est lancé avec frénésie dans un tour de France des élus locaux, ne comptant plus son temps, prenant force notes et découvrant enfin les vertus de la proximité. En même temps », il n'avait pas le choix, parce que c'est aux fantassins de la République, aux élus eux-mêmes qu'il faut redonner confiance, et ce maintenant. Il est indispensable de leur apporter l'appui de la Nation qu'ils incarnent au quotidien auprès de nos concitoyens, leur signifier que la confiance des Français, dont plus de 80 % ont une image positive de leur maire, se traduit en actes, en clair qu'on ne les laisse pas tomber. pour atteindre cet objectif que le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique nous est présenté aujourd'hui ? D'un naturel optimiste, je me plais à le croire. Car oui, la situation est devenue intenable pour les élus locaux, les maires en tête. Entre sentiment d'abandon et absence de reconnaissance, ces derniers ont exprimé récemment un sentiment d'usure et d'impuissance encore jamais éprouvé Au Sénat, conformément à la responsabilité que nous confère l'article 24 de la Constitution, nous avions entendu de longue date les appels au secours montant des territoires. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui reprend d'ailleurs un grand nombre des positions tenues par le Sénat depuis plusieurs années, notamment sur l'articulation communes-EPCI ou encore sur les conditions d'exercice des mandats. Il était plus qu'urgent d'agir Apportant la preuve tangible que la vision du Sénat n'est pas « datée », sous l'impulsion de son président Philippe Bas, que je veux ici saluer, la commission des lois a lancé, de manière inédite, une vaste consultation des maires, des adjoints et des conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonctions. Les résultats n'ont pas tardé à remonter du terrain, en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. La commission des lois a donc logiquement pris en compte leurs justes demandes et amendé profondément le projet de loi Engagement et proximité. sur lesquels le texte initial avait été jugé timoré ou frileux par les associations d'élus, nous avons ajouté des dispositions nettement plus ambitieuses.

C'est ainsi que nous avons entendu le souhait mille fois répété des associations d'élus de voir supprimer purement et simplement le transfert obligatoire de la compétence en matière d'eau et d'assainissement dans les communautés de communes et d'agglomération. Il ne s'agit plus là du mécanisme limité et compliqué proposé au travers du texte initial, mais d'une solution simple et efficace. En ce qui concerne le renforcement des pouvoirs de police du maire, nous proposons notamment d'augmenter fortement le montant des amendes pouvant accompagner une astreinte et de codifier la possibilité d'interdire la vente de boissons alcoolisées la nuit dans les communes. C'est à nous qu'il revient de faire en sorte que des orientations fermes de politique pénale en cas d'agression d'élus locaux soient diffusées à l'ensemble des parquets. C'est à nous de faire en sorte que les conditions de mutualisation des polices municipales soient assouplies. Mes chers collègues, chacun d'entre nous le sait personnellement, la vie politique est ardue, chronophage et souvent ingrate. Mais chacun d'entre nous sait aussi qu'elle offre toutes les richesses d'un engagement humain au service de l'intérêt général, d'un projet de territoire, d'une Nation.

Mon département abrite la plus grande communauté d'agglomération de France par le nombre de communes membres : 158, pour 238 conseillers communautaires.

Certes, dans un cas comme dans l'autre, c'est la volonté des élus qui s'est exprimée, à de larges majorités : en Pays basque, elle était le puissant écho d'une volonté d'existence institutionnelle ; en Béarn, c'est l'esprit montagnard et « valléen » qui s'est manifesté. Au-delà de ces contingences locales, ces exemples démontrent que le découpage intercommunal recouvre aujourd'hui des réalités bien différentes. Or la législation n'a jamais été adaptée à cette diversité des situations. En effet, sous le quinquennat précédent, deux courbes ont été prolongées sans jamais qu'elles se rencontrent, avec, d'une part, le meccano institutionnel de la loi NOTRe, qui fut tout sauf l'acte III de la décentralisation, cher Éric Kerrouche, et, d'autre part, l'énergie déployée par les préfets pour établir de vastes intercommunalités, parfois en recourant au « passer outre », c'est-à-dire en passant outre la volonté des élus. Pourtant, en 1981, Gaston Defferre soulignait que « c'est bien servir la France que de permettre aux élus de décider sur place des solutions à apporter aux problèmes qu'ils connaissent mieux que quiconque A-t-on continué dans cette voie au cours des dernières années ? Hélas, non ! Bien au contraire, la tentation recentralisatrice a pris le dessus.

Sénat. Ce texte ne règle pas tout, mais il recherche, pour la première fois depuis longtemps, un nouvel équilibre entre la commune et l'intercommunalité. Il vise à une meilleure participation des maires à la gouvernance des intercommunalités, renouant ainsi avec une vision essentielle : la commune est le premier lieu où se vit la démocratie. L'intercommunalité relève d'une dynamique territoriale,

pourrait être l'occasion d'aller plus loin en mariant, dans les intercommunalités « XXL », cohérence des politiques publiques à grande échelle et proximité dans la gestion grâce aux pôles territoriaux. Enfin, en bon girondin et élu du Pays basque que je suis, j'avoue aussi attendre de votre texte un nouvel et réel acte de décentralisation d'une volonté sincère d'installer solidement dans notre pays le droit à la différenciation. Je dois le dire, cette attente forte a été largement refroidie par le discours du Premier ministre à Bordeaux.

l'EPCI est un établissement public au service de ses adhérents que sont les communes. L'ensemble forme le bloc communal,

sans aucun doute depuis un an sous le régime d'une loi qui aurait supprimé les irritants de la loi NOTRe, qui semblent aujourd'hui vous donner tant d'urticaire

dans l'aménagement des dispositions applicables aux collectivités territoriales, concernant notamment la relation entre l'intercommunalité et ses communes membres.

la répartition des compétences entre les communes et l'intercommunalité, avec la fin des compétences optionnelles, vous n'en voulez pas ; la disposition qui vise à neutraliser les effets d'un retour de compétences aux communes sur le montant total des dotations d'intercommunalité, vous n'en voulez pas

à son conseil municipal un triplement de son indemnité à la charge de la commune. Très bien ! Quant aux pouvoirs du maire, je vous sais gré d'avoir ajouté dans votre propre texte, une lettre rectificative, quelques dispositions à celles qui y figuraient initialement. Je serais heureux que vous acceptiez les propositions que nous avons formulées et d'ores et déjà intégrées au texte de la commission des lois pour renforcer

que les maires soient confortés par rapport à toutes ces incivilités et à toutes ces violences qui aujourd'hui accablent certains d'entre eux. a eu deux ans, monsieur le ministre, pour réfléchir. Vous nous demandez une année supplémentaire pour franchir une étape dans le développement des libertés locales, en invoquant toute la difficulté technique qu'il y aura à poser de nouvelles règles pour les départements et les régions. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts. J'ai déposé avec Mathieu Darnaud et Bruno Retailleau des textes, prévoyant même un socle constitutionnel. Nous souhaitons pouvoir en débattre très rapidement. Pourquoi vous faut-il tant de temps pour réfléchir alors que la question des libertés locales est aujourd'hui cruciale, comme vous l'avez vous-même expliqué il y a un instant ?

à la coordination du bloc départemental, du bloc régional et du bloc communal, ce n'est pas trop. Je crois d'ailleurs savoir que, même au sein de cet hémicycle, le débat n'a pas encore eu lieu, puisque

de le protéger. La loi NOTRe a déjà retiré la clause de compétence générale aux départements et transféré un grand nombre de leurs compétences aux régions, notamment en matière de transport et de développement économique. Les élus s'inquiètent à juste titre de la future réforme de la fiscalité locale, qui portera un nouveau coup dur aux départements et à leur autonomie. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d'ôter aux départements leur dernier levier en matière de fiscalité locale, la taxe sur le foncier non bâti,

à la loi NOTRe, certains vantant ses mérites, d'autres dénonçant ses effets néfastes pour nos collectivités.

à l'abroger. Cette loi marque le paroxysme des politiques menées depuis la fin du XX siècle, et plus particulièrement ces dernières années, en matière de décentralisation,

qui leur tenaient pourtant à coeur et dont elles pouvaient assurer le bon exercice. Dans le même temps, cette loi a révélé un désir de réduire, progressivement mais sûrement, la place des départements, qui ont perdu leur clause de compétence générale et vu nombre de leurs compétences passer aux mains des régions. Les gouvernements successifs menant ces politiques ne rêvent que de grandes régions européennes et de métropoles. Aux contours naturels des territoires se sont substitués

il est quelque peu disruptif ... On reconnaît bien là l'audace des sénateurs, parfois sous-estimée ! Cet amendement vise à demander l'abrogation

comment ont pu apparaître ces fameux irritants, qui ne sont pas simplement issus de la loi NOTRe. Il conviendrait également de savoir ce que ces politiques ont apporté aux citoyens, aux élus, aux collectivités et à la République. À l'heure où le Gouvernement souhaite rationaliser les services publics en coupant dans les moyens et dans les effectifs,

Il en existe déjà dans de nombreux EPCI. Ces instances ont un objet d'intérêt général, à savoir conforter la place des maires au sein des EPCI, notamment lorsqu'ils ne sont pas membres du bureau. Trop souvent en effet, les maires des petites communes ont des difficultés à se faire entendre au sein des intercommunalités. Par ailleurs, créer une telle instance de dialogue et de concertation entre les exécutifs locaux sur des projets communautaires, ainsi que sur des questions de coordination entre les actions engagées par les communes et celles des EPCI, constituerait

eux. Faut-il rendre obligatoire la mise en place d'une telle conférence des maires, sorte de bureau élargi, avec le risque d'alourdir la réglementation et d'imposer de nouvelles contraintes ? Doit-on, au contraire, la rendre facultative ? Dans certains cas, elle ne verra alors pas le jour, l'exécutif intercommunal pouvant n'avoir aucun désir de voir se réunir régulièrement l'ensemble des maires. des maires. Faut-il opter pour un dispositif facultatif, mais en donnant la possibilité, par exemple à 30 % des maires de l'EPCI, d'imposer la création d'une telle instance de dialogue,

ne se sentent pas suffisamment associés à la gouvernance des EPCI. Nous avons donc formulé douze recommandations visant à renforcer la place des élus municipaux dans cette gouvernance. La première d'entre elles est ainsi intitulée : « se doter d'une charte de gouvernance pour définir les rôles respectifs entre les communes et la communauté, et formaliser la coopération entre communes membres dans le respect de chaque territoire ». encore la proposition n° 4 : « prévoir, dans le fonctionnement de l'EPCI, une instance spécifique de dialogue des maires et faire en sorte que ceux-ci deviennent des relais de l'action communautaire dans chaque territoire ». Ces recommandations sont reprises au travers de l'article 1 du présent projet de loi, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela témoigne d'une belle concordance de nos préoccupations

de rencontres organisées sur le territoire avec les élus locaux, nous avons constaté que persistait un sentiment de frustration, dû notamment à un manque de débat tenant soit au nombre

Ils constituent la première marche de la démocratie dans notre pays, ils mettent en oeuvre des projets d'aménagement, ils sont les animateurs infatigables de leur commune, ils donnent une portée concrète à un premier niveau de solidarité. Je veux me faire ici l'écho de leurs difficultés, mais aussi de leur volonté de construire, encore et toujours, un avenir possible sur des territoires économiquement et socialement éprouvés.

du temps à titre quasiment bénévole, l'engagement du maire est synonyme de sacrifices personnels. Son coût humain est important en termes de responsabilité, d'exposition à la violence, de normes à appréhender, de vie familiale perturbée, de compatibilité avec un exercice professionnel. Évolution ou suppression des services publics, extension souvent à marche forcée des périmètres des intercommunalités amenant à s'interroger sur la nature des processus démocratiques qui se déroulent en leur sein, dévitalisation des centres-bourgs ou centres-villes, concentration de familles en grande souffrance : les élus locaux sont confrontés à des problématiques qui dépassent leur pouvoir d'action, mais dont les effets les touchent directement.

l'autorité, l'initiative du maire demeurent indispensables à une vie équilibrée dans la ruralité de notre pays. Vous l'aurez compris, je soutiendrai la création

Nous sommes donc en présence d'EPCI pouvant compter quarante, voire soixante communes membres, et à cheval sur deux départements, parfois même sur deux régions. Le périmètre d'action des intercommunalités rurales et de montagne renforce, à n'en pas douter, le sentiment d'éloignement et de disparition des communes membres dans des ensembles dont l'identité est en construction. Dans ce contexte, le transfert de compétences complet et le transfert de compétences morcelé, quand il s'agit par exemple de la compétence scolaire ou de l'urbanisme, sont largement vécus comme une dépossession par les maires des petites communes. La création de la conférence des maires est une bonne chose. Pour autant, à notre sens, elle n'est pas suffisante. Pierre Mendès France écrivait, dans que « la démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen non seulement sur les affaires de l'État, mais sur celles de la région, de la commune, de la coopérative, de l'association, de la profession. » Il en va de même pour les maires de petites communes membres de grandes communautés de communes. Nous pensons qu'il faut inventer un autre mode de gouvernance, associant de manière plus continue les maires. Ce texte, de manière générale, tend à renforcer le rôle institutionnel des maires, en améliorant la communication et en renforçant les possibilités de blocage d'un projet. C'est une étape à prendre en compte. Il faudrait, en parallèle, veiller à améliorer le rôle décisionnel des communes et mettre en place une véritable codécision, un travail en commun. Notre groupe présentera plusieurs amendements

on a en effet réussi le tour de force de fragiliser les communes comme échelons de proximité et d'affaiblir l'idée intercommunale au profit d'une supracommunalité ivre d'elle-même et portée par une logique d'intégration à marche forcée. Ce double mouvement, à l'oeuvre depuis quelques années, a profondément bouleversé l'équilibre au sein du bloc communal et nourri des tensions très dommageables dans le couple communes-communauté de communes. Cette situation conduit aujourd'hui le Gouvernement- sur la requête, il est vrai, du Sénat -à tenter de réformer et de répondre à un besoin de proximité de plus en plus fort issu des territoires,

Vous pouvez compter sur le Sénat et sa commission des lois pour renforcer les mesures proposées par le Gouvernement, pour peu, évidemment, qu'elles visent à consolider la place des communes et des maires dans le fonctionnement de l'intercommunalité. de cet article, qui prévoit l'instauration d'un pacte de gouvernance. Seule une véritable association des maires à la gouvernance de l'intercommunalité permettra de trouver un équilibre entre les communes, dont l'intercommunalité est en principe l'émanation.

et la connaissance des problématiques communes et, finalement, de faire en sorte que la commune redevienne, comme l'a dit notre collègue Mathieu Darnaud, la porte d'entrée de l'intercommunalité. La parole est à M. Maurice Antiste,

a ainsi été élaboré à la suite de rencontres avec les associations d'élus, les parlementaires engagés sur le sujet des collectivités territoriales et les présidents de groupe du Sénat. Plus de 500 contributions ont ainsi été reçues, analysées et intégrées. L'exécutif ne nous avait pas habitués à tant d'égards ! Il faut dire que les maires et, plus généralement, les 600 000 élus locaux, se sentant dépossédés, déclassés et impuissants, ont fait entendre leurs doléances pendant le grand débat national. L'objectif annoncé de « revaloriser le bloc communal et la figure du maire, qui est centrale dans notre histoire et notre identité commune »- je reprends ici vos propos, monsieur le ministre -ne peut trouver qu'un écho favorable en ce lieu. Ce texte entend valoriser et accompagner ceux qui s'engagent pour la collectivité, en améliorant les conditions d'exercice des mandats locaux. Il vise également à étendre les libertés locales, conforter le rôle du maire pour que celui-ci puisse trouver un meilleur équilibre avec son intercommunalité, à simplifier le quotidien des élus locaux et à mieux adapter certaines règles ou certains seuils aux réalités territoriales. de loi va effectivement dans le bon sens, ses mesures, par ailleurs hétéroclites, seront-elles suffisantes pour atténuer le mal-être des maires, dont près de la moitié sont prêts à jeter l'éponge à l'occasion du prochain scrutin municipal de mars 2020 ? Elles constituent plutôt, à mon sens, une avancée, un premier pas qui doit en amener d'autres ! Il y a urgence à revaloriser, à revitaliser la démocratie en agissant au plus près des territoires. Cela devrait également passer, et c'est ce qui manque aussi à ce texte,

la relation des maires avec une intercommunalité qui compte 158 communes et 238 conseillers communautaires passe obligatoirement aussi par des pôles territoriaux. Les maires ont besoin, dans ces grands ensembles qu'ils ont

Je les comprends, car une intercommunalité ne peut convenablement fonctionner si elle n'est pas, d'une certaine manière, « partagée ». J'aurais d'ailleurs pu dire la même chose au sujet du pacte de gouvernance.

Rappelons que cette instance aura pour objet de débattre des orientations politiques et des décisions importantes de l'EPCI. En rendant obligatoire, et non plus facultative, la mise en place d'un tel outil, on assurerait à toutes les petites communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux. C'est très important ; elles ne sont pas des communes de seconde zone ! Le Gouvernement, par la voix du Premier ministre, n'a-t-il pas récemment présenté un « agenda rural » Il faut passer de la parole aux actes : au sein des intercommunalités, tout doit être fait pour garantir l'équilibre territorial, le respect de la souveraineté des communes, la recherche du plus large consensus et le partage des décisions. de la conférence des maires obligatoire, on reconnaîtra le rôle central des maires. Il me semble que telle est l'ambition de ce texte.

autant que faire se peut le texte, voire nous accorder sur certaines dispositions. En l'espèce, j'ai du mal à comprendre ce qui empêche de faire du pacte de gouvernance la règle de droit commun

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que les éléments bénéfiques de ce pacte puissent profiter à toutes les communes de France.

est en effet essentiel au bon fonctionnement d'un EPCI. Il permet d'établir des relations satisfaisantes avec les communes et leurs élus. L'établissement d'un pacte de gouvernance est, d'ores et déjà, une pratique courante, et le présent dispositif reprend largement ce qui existe dans nombre d'EPCI. Tout en respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales, nous estimons que donner à ce pacte un caractère facultatif n'encouragera pas les EPCI au sein desquels

Rendre obligatoire ce pacte permettra de poser un cadre consensuel de réflexion sur la gouvernance de l'intercommunalité et les relations avec les communes membres. À chaque renouvellement ou création d'un EPCI, il semble cohérent de partir sur de bonnes bases en ouvrant ce débat entre les communes et en leur laissant ensuite la possibilité ensuite de définir ce pacte comme elles le souhaitent, en coordination avec l'EPCI.

vise à rendre obligatoire l'adoption d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'EPCI dans les neuf mois suivant la mise en place du conseil communautaire.

L'étude d'impact du projet de loi indique que les métropoles sont des EPCI très intégrés. Le présent article prévoit ainsi l'obligation de créer une conférence des maires pour les métropoles, en remplacement de l'actuelle conférence métropolitaine.

est à M. Maurice Antiste. Il s'agit d'un amendement de repli, dans l'hypothèse où les conseils de développement deviendraient facultatifs. Les conseils de développement sont en cours de généralisation dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Cette dynamique est récente et fragile. Pour perdurer, elle a encore besoin d'être encouragée et accompagnée, jusqu'à assurer un maillage suffisant dans l'ensemble des territoires, ruraux et urbains. Ne pas favoriser l'existence des conseils de développement briserait l'élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne, fragilisant les plus récents d'entre eux dans un contexte de renouvellement des mandats. Il y a lieu de prendre en compte les apports des conseils de développement. Outre leur contribution à l'enrichissement des politiques publiques, ils constituent, à l'échelle intercommunale, l'un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s'exprimer de manière argumentée et se réduire de façon apaisée. Dans un contexte marqué par la défiance et l'urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d'écoute et de respect de l'autre, d'attention à l'intérêt général et d'une citoyenneté active et responsable. Il est donc nécessaire,

parole est à M. Henri Leroy. Le pacte de gouvernance est un outil important, qui permet aux élus locaux, et surtout à l'exécutif de chaque commune membre, de s'accorder sur le fonctionnement de leur EPCI, ainsi que sur l'ordre du jour

en disposant que le pacte de gouvernance prévoie, le cas échéant, l'établissement de liens avec les collectivités voisines.

Ainsi, pour pleinement satisfaire l'ensemble des communes et des administrés d'un EPCI, il peut être nécessaire d'envisager des partenariats avec les collectivités voisines, en l'absence de pôles

sous un autre angle, celui du regard de nos concitoyens, les habitudes de vie de ceux-ci dépassent souvent le cadre administratif de leur EPCI de résidence. Aussi, même avec des EPCI agrandis, il s'agit d'anticiper le fait que ces continuités s'épanouiront et que des connexions seront tentées, voire établies. En présence d'un PETR, PETR, qui a pour objet partiel de répondre à cette logique, l'EPCI en périphérie de ce PETR visera à s'assurer des continuités hors PETR pour certaines

précédente. Afin de permettre une meilleure lisibilité des documents qui ont trait au fonctionnement interne de l'EPCI, je vous propose, mes chers collègues, d'inscrire dans la loi que le pacte de gouvernance doit être annexé au règlement intérieur des EPCI.

au coeur du village républicain, si je puis dire. Un élément extrêmement important doit être pris en considération : la discussion portant sur l'élaboration ou non d'un pacte de gouvernance est obligatoire,

qu'il y avait presque autant d'EPCI que de réalités territoriales et de réalités de gouvernance. Tout EPCI peut compléter le pacte de gouvernance à sa guise, en y ajoutant des éléments qui relèvent même du règlement intérieur. Ce pacte peut donc être enrichi selon les choix et la volonté des élus locaux.

nous avons proposé à M. Joly d'émettre un avis favorable à son amendement sous réserve qu'il rectifie ce dernier, en prévoyant que le pacte de gouvernance

que les assemblées délibératives, en clair le conseil communautaire et les commissions ; le pacte de gouvernance, lui, peut aller au-delà, notamment avec les questions de représentation et de délégation - on y reviendra à propos d'autres articles du projet de loi.

technique ! ... me semble quelque peu léger par rapport à l'enjeu du pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, c'est un projet politique et un projet de territoire. Il me semble que s'engager à réaliser un tel document dans un délai de six mois est une gageure, qui va mettre les élus en difficulté. On l'a bien dit, l'intercommunalité est un espace de consensus et d'élaboration de projets collectifs.

des difficultés à comprendre les blocages des rapporteurs, d'autant que je viens d'écouter attentivement attentivement Mme Gatel, qui nous explique que le pacte de gouvernance devait être un projet politique et un projet de territoire

services, et évidemment des données financières. On sait en effet qu'il y a une interaction très forte entre les choix financiers réalisés par l'intercommunalité et les dotations ou les finances des communes.

et de confirmer cette volonté de donner plus de liberté aux acteurs des collectivités locales. Vous ne diriez

mais il ne nous semble pas forcément pertinent de rendre cette démarche obligatoire par la loi, sachant que les adhésions à des espaces plus vastes relèvent de délibérations prises par le conseil communautaire, et parfois même